La parole est d'abord Madame Jocelyne Guidez pour une mise au point au sujet d'un vote, vous avez la parole cher collègue. Oui merci monsieur le président, madame ma collègue Christine Herzog sénatrice de la Moselle souhaite modifier son vote du scrutin numéro 29 sur l'ensemble du projet de loi relative à à l'accélération de la production d'énergie renouvelables du samedi 4 novembre 2022 en ne prenant pas part au vote, au lieu de son vote pour merci. Acte est donné de votre mise au point, elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l'analyse politique du scrutin concernés. Madame la ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale, en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour 2023 dans la discussion générale, la parole est à monsieur François Braun Ministre de la santé et la prévention, vous avez la parole monsieur le Ministre. Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires sociales. Madame, monsieur les ministres, madame la rapporteure générale, mesdames, messieurs les rapporteurs mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs. C'est un avec engagement confiance détermination que je viens débattre dans cet hémicycle pour l'examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023. Dans le titre même de ce projet de loi il y a sécurité cette sécurité, nous la devons d'abord à nos concitoyens pour qu'ils puissent accéder facilement à la santé, d'où qu'ils viennent et quelle que soit leur situation. L'universalité de l'accès à la santé, c'est mon moteur, c'est mon engagement : l'engagement de mon action en tant que ministre. Cette sécurité, nous la devons aussi à ce même système de santé qui se met chaque jour au chevet des Françaises et des Français en ville comme à l'hôpital avec abnégation et dans des conditions que je c'est difficile. Prendre soin de ceux qui prennent soin de nous, c'est une de mes priorités en tant que ministre de la Santé et de la prévention, c'est tout l'engagement de ce gouvernement et de cette majorité. Avec ce Plfss nous faisons le choix d'un système de santé renforcée et plus juste pour mieux répondre aux besoins de nos concitoyens et de nos professionnels. Alors concrètement comment se traduit cette ambition, elle passe d'apport par un investissement en rapport avec les enjeux de la santé. Pour 2023, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, l'Ondam est proposé à un niveau historique de plus 3 7 % hors dépenses de crise sanitaire, c'est important de le redire. Cette augmentation s'inscrit dans la droite ligne de l'effort d'investissement que nous avons réalisé ces dernières années, notamment avec le Ségur de la santé. Au delà de cet investissement soutenu le PLFSS porte aussi des mesures fortes. Notre ambition, c'est avant tout d'offrir à nos concitoyens, un pays où chacun peut accéder facilement aux soins, peu importe l'endroit où il vit, où ses revenus. C'est pour cette raison que nous menons avec ce Plfss une lutte déterminée contre toutes les inégalités d'accès à la santé territoriale financière sociétal. C'est tout simplement un enjeu de justice sociale, à l'heure où près de 4 millions de Français vivent dans un territoire sous-doté et où 6 millions de nos concitoyens n'ont pas de médecin traitant. Cette situation elle tient à l'effet des décisions passées qui nous conduisent à enregistré aujourd'hui un système de santé à bout de souffle, avec en particulier une baisse sans précédent de nos ressources, notamment médicale. Pour faire face, nous devons agir sur tous les. Pour mieux inciter les professionnels de santé à s'installer dans les zones sous-dotées ce PLFSS vise à renforcer l'impact des aides à l'installation. Ces aides sont complexes, elles sont multiples, elles sont mal connues et mal comprise des professionnels qui ne s'y retrouve plus. Nous proposons donc de les simplifier. Nous avons aussi un enjeu important à mieux accompagner les médecins proches de la retraite pour qu'ils poursuivent leur activité, de même qu'à faire revenir des médecins retraités actifs qui en aurait l'envie. Le président de la République l'a annoncé, c'est une mesure forte face aux territoires sous-dotés, nous exonère auront de cotisations retraite les médecins retraités qui souhaiteraient prolonger ou reprendre leur engagement au service de nos concitoyens. Aussi, à l'heure où s'ouvrent les négociations conventionnelles, nous proposons de créer un cadre plus adapté pour que ces dernières soient pleinement fondée sur la logique d'engagements réciproques, particulièrement vis-à-vis des territoires et de la permanence des soins. Enfin, et je sais le soutien de cette assemblée, nous formerons aussi mieux les futurs médecins généralistes, notamment pour mieux les préparer à une installation plus rapide en sortie d'études grâce à la 4ème année d'internat. Si celle-ci a pleinement vocation à se faire en ambulatoire, j'ai entendu que dans quelques situations très ciblée exceptionnel, il était important pour les étudiants de pouvoir déroger à ce principe. Le gouvernement a déposé un amendement en ce sens pour tenir compte des échanges au cours en cours dans le cadre de la mission sur les conditions de mise en oeuvre de cette 4ème année. Enfin, je tiens à le redire, si nous favoriserons cet exercice en zone sous-dense, ce ne sera pas une obligation. Ce PLFSS a aussi pour ambition de renforcer notre hôpital avec des moyens et une reconnaissance à la hauteur du service qu'il rend aux Français. Trop longtemps non soignants ont dû mettre les bouchées doubles pour compenser des décennies d'économies réalisées sur l'hôpital, au prix d'un désespoir grandissant chez certains de nos professionnels. Ce sont ces choix passés répétées qui font que nous avons aujourd'hui à gérer des urgences successives. J'étais par exemple avec les représentants du secteur de pédiatrie, la semaine dernière pour mettre en place des mesures rapides face à une épidémie de bronchiolite précoce qui fait peser une pression accrue sur des services déjà fragilisé. Si j'assume totalement de devoir gérer des situations de tension j'assume aussi d'accélérer les transformations plus profondes, structurelles qui, seules, nous permettront de retrouver de la sérénité de la confiance en l'avenir et de l'excellence pour notre hôpital. J'ai notamment la conviction qu'il est temps de régler cette question de l'intérim, qui lorsqu'il devient mercenaire est un poison pour nos équipes et la stabilité de nos établissements. Ce Plfss prévoit ainsi de ne pas autoriser cette pratique de l'intérim, en début de carrière. C'est bon pour les hôpitaux, c'est sécurisant pour les jeunes professionnels. Au total, le soutien à l'hôpital se traduit par un Ondam hospitalier qui progresse de 4 virgule un pour 100. C'est un effort de plus de 100 milliards d'euros, en augmentation de 3 6 milliards d'euros par rapport à 2022. Les travaux sont par ailleurs en cours pour la rectification de l'Ondam 2022 dans la suite des annonces récentes de soutien à l'hôpital pour l'hiver, et notamment la prolongation de majoration de nuit d'ici la mise en oeuvre de travaux plus structurelle. Et ceci en maintenant aussi notre effort sur les soins de ville à l'aube de l'ouverture des négociations conventionnelles avec les médecins libéraux. Le choix de ce Plfss cette enfin d'offrir à nos concitoyens, un pays où les maladies sont prévenus avant d'être soigné. C'est une clé essentielle de l'avenir de notre santé, j'en ai aussi la conviction profonde. Oui, avec ce texte, nous faisons un grand pas en avant pour prendre la prévention bien réelle et présente dans notre société. Ma philosophie, c'est de donner toutes les clés à nos concitoyens pour prendre soin de leur santé en sortant des messages de culpabilisation en rendant la prévention attractive. Nous proposons ainsi de mettre en place des rendez vous de prévention qui prendront la forme de bilan de santé aux âges clés de la vie, pris en charge à 100 % par l'assurance maladie. Cette mesure a de vocation, d'une part, aller chercher les patients les plus éloignées du système de santé qui ne voit pas souvent leur médecin et d'autre part, agir sur la durée, en proposant des parcours de santé autour de ces rendez-vous permettant d'éviter des maladies et de mieux prendre en compte des enjeux essentiels comme la santé mentale, la santé des femmes, la prévention des cancers. le gouvernement s'engage également dans ce PLFSS pour la santé sexuelle et pour la santé des femmes à travers des mesures concrètes, nous proposons ainsi d'élargir à d'autres infections sexuellement transmissibles que le VIH, le dépistage sans ordonnance et gratuit, pris en charge à 100 % pour les moins de 26 ans. Par ailleurs, alors que seulement 10 % des contraceptions d'urgence sont remboursés actuellement nous voulons élargir la délivrance gratuite de la contraception d'urgence pour toutes les femmes, peu importe l'orage. Enfin, la crise sanitaire récente a montré à quel point se faire vacciner est essentielle pour se protéger et protéger les autres. Nous proposons donc d'élargir la prescription et la réalisation de vaccins ou pharmaciens, sages-femmes et infirmiers, ce qui est d'autant plus essentiel que nous lançons actuellement une campagne de vaccination à la fois contre la grippe et le Covid 19. Nous avons souhaité à ce titre, conserver à l'issue des débats à l'Assemblée nationale, les amendements prévoyant d'autoriser les étudiants en 3ème cycle de médecine et en pharmacie à vacciner. En un mot ce PLFSS concrétise notre ambition de faire rapidement de la prévention un pilier à part entière de notre système de santé. Ce PLFSS est enfin un texte de responsabilité qui tient compte de l'enjeu majeur de soutenabilité de notre système de santé. J'assume le fait que ce redressement sera fait par le renforcement de la pertinence et de la qualité de la réponse aux besoins de santé. Nous travaillerons d'ailleurs aussi dans le cadre du Conseil national de la refondation santé sur ce pacte de soutenabilité à faire avec les Français et tous les professionnels. D'ores et déjà ce budget de la Sécurité sociale, propose des mesures que nous pensions juste et proportionnée pour que nos déficits ne pèse pas sur les générations futures et que nous ne soyons pas amenés à baisser les droits ni à augmenter les impôts, comme s'y est engagé le gouvernement. Nous allons ainsi exiger du secteur de la radiologie qui renforce la transparence et l'information sur le coût de ces équipements matériels. Nous allons ainsi exigé, nous allons également pardon demandé une contribution à la biologie, en ouvrant une négociation avec ce secteur parallèlement à l'engagement d'une mission pour mieux préparer son avenir. Nous allons aussi réguler la trajectoire très dynamique de dépenses sur les médicaments. Tout en préservant les engagements pris pour soutenir nos capacités d'innovation, de production de nos plus vieux médicaments qui restent nécessaires dans le quotidien des Français, et notre souveraineté nationale et européenne. Nous travaillerons également avec les complémentaires santé sur de multiples chantiers notamment pour élaborer un partage équitable des remboursements dans le Champ de la santé. Enfin, ce Plfss adresse aussi un message de fermeté à l'égard de tous les types de fraudes. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, vous le voyez, notre ambition pour la santé de nos concitoyens 50 pleinement dans le PLFSS que je vous présente aujourd'hui. Notre engagement pour la santé des Françaises et des Français n'est pas fait de mot, il est fait de moyens de propositions nouvelles et de réformes courageuses. Ce PLFSS pour l'année 2023 7 c'est une première Pierre à l'effort de refondation que nous voulons mener pour que la devise de notre République : liberté, égalité, fraternité, soit une réalité en matière de santé comme dans tous les autres aspects de la vie de nos concitoyens. Je le dis aussi avec franchise ce PLFSS c'est une première page, une page importante, mais il n'achète pas l'ensemble des réponses que nous devons à nos concitoyens. Cela sera notamment le rôle des négociations conventionnelles pour lesquels j'ai rendu public mes orientations, il y a quelques jours, et celui du Conseil national de la refondation lance en santé que j'ai lancé le mois dernier au Mans et qui crée une dynamique importante dans les territoires en lien, principalement avec les élus. Bien sûr, ces travaux n'ont pas vocation à remplacer le débat au sein de la représentation nationale, ils en sont complémentaires. Malgré le contexte, le débat fut fécond à l'Assemblée nationale. Nous avons pu en lien avec les députés de l'arc républicain progresser sur des sujets importants comme le cumul emploi-retraite des médecins le contenu des rendez vous de prévention, l'encadrement de la 4ème année d'internat de médecine générale ou la permanence des soins. Nous avons pu également progresser sur la mise en place d'expérimentation sur le dépistage de la drépanocytose ou la réalisation de certificat de décès par les infirmières par exemple. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, construisons ensemble des apports utile au service des Français, je vous remercie. Merci. Le ministre. La parole est maintenant monsieur Jean-Christophe Combe Ministre des Solidarités de l'Autonomie et des Personnes handicapées, vous avez la parole monsieur le Ministre. Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure générale de la commission des affaires sociales, mesdames et messieurs les rapporteurs mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, en ouvrant avec vous la discussion du budget de la Sécurité sociale pour 2023 je veux avoir une pensée pour tous les professionnels du soin pour tous les professionnels du lien qui, cette année encore, ont accompagné nos compatriotes malgré la crise, malgré les doutes et malgré la pression. L'épidémie de Covid les têtes canicule, le manque de personnel sur tous les bancs, nous connaissons la situation et sur tous les bancs, nous saluons le rôle décisif de ces femmes et de ces hommes. En cette période de difficultés et d'incertitudes, le choix que nous vous proposons pour l'année prochaine et d'augmenter les moyens que la nation consacre aux personnes âgées en perte d'autonomie aux personnes en situation de handicap et aux familles

cela marque aussi la volonté du gouvernement de protéger les Français qui en ont le plus besoin, tout en poursuivant la réforme de notre modèle social pour qu'il soit plus performant ces 3 milliards d'euros supplémentaires, nous proposons de les engager pour régler des problèmes du quotidien, restaurer la confiance dans les EPHAD et augmenter le nombre de soignants pour que les enfants ne s'inquiète pas pour leurs parents âgés et que nos aînés soient dignement accompagner, soutenir les services à domicile pour que chacun puisse avoir le choix de rester chez soi et dit bien vieillir, faciliter l'accès à des solutions d'accueil pour les jeunes enfants, pour permettre à leurs parents, de travailler, je pense notamment aux femmes et aux familles monoparentales ou encore pouvoir scolariser dans de bonnes conditions, son enfant en situation de handicap, voilà quelques exemples de sujets sur lesquels ce budget va nous permettre d'avancer ces 3 milliards d'euros supplémentaires sont aussi là pour protéger de l'inflation, le secteur médico-social déjà fragilisée par les tensions de recrutement, nous faisons par exemple le choix de compenser l'impact de l'inflation sur les charges non salariales des dotations de soins, des Ephad et de faire bénéficier ces établissements du bouclier tarifaire de l'énergie ce secteur économique est précieux en termes d'emploi est indispensable en matière de service pour un grand nombre de Français nous assumons donc ce soutien qui est d'intérêt général, ce soutien à la consolidation du secteur, nous le faisons face à l'urgence, mais nous le faisons également dans la durée avec la CNSA et avec l'ensemble des acteurs, ce budget est un nouveau signe fort de la volonté de l'État. La question des moyens est importante, mais celle de la méthode l'est tout autant, et pour cela je fait clairement le choix du dialogue avec les secteurs concernés et de la co-construction avec les collectivités, notamment avec les départements, j'étais ce matin avec les aidants, je serai demain avec les assistantes maternelles, j'étais en fin de semaine dans la Marne, avec les élus et tous les acteurs du grand âge, toujours dans cet esprit d'écoute et de recherche de solutions car les solutions ne peuvent pas attendre, c'est notamment le cas en matière d'autonomie, je le disais, nous devons restaurer la confiance dans les EPHAD et cela passe notamment par davantage de contrôle et de sanction sur ce sujet, nous nous sommes appuyés sur les travaux parlementaires et je salue la sénatrice Michèle Meunier et le sénateur Bernard Bonne, coauteur d'un rapport dont de nombreuses recommandations ont déjà été reprises et dont d'autres se retrouvent dans ce texte, l'article 32 renforcée par l'Assemblée Nationale nous permettra ainsi de renforcer le contrôle et de durcir les sanctions contre les établissements fautifs, je pense aussi au financement des moyens humains pour contrôler 100 % des établissements dans les deux ans comme nous l'avons annoncé ces contrôles ont déjà commencé, j'en rendrai compte régulièrement et en toute transparence, devant la représentation nationale, cette transparence, nous la devons aux familles et aux professionnels eux-mêmes, restaurer la confiance dans les EPHAD c'est aussi soutenir leur professionnel, notre objectif est clair : 50000 soignants de plus dans les prochaines années et 3000 dès 2023, j'entends les critiques de celles et ceux qui considèrent que nous n'allons pas assez vite, mais j'étais il y a encore quelques semaines, directeur général de la Croix-Rouge française et c'est précisément parce que je connais la réalité de la situation que je veux tenir devant vous un discours de vérité, ce serait bien trop facile de promettre des centaines de milliers de postes si nous ne sommes pas capables de former, d'attirer et de fidéliser les professionnels, c'est donc bien sûr l'ensemble du problème que nous agissons, il y a la question de la rémunération sur laquelle aucune majorité n'a, n'a fait autant que la nôtre mais aussi regarder les questions de formation de management de parcours de reconnaissance et de santé de nos professionnels dans la droite ligne de la loi de financement pour 2022, le gouvernement propose de poursuivre et d'accélérer sur le développement du domicile d'abord en renforçant les services de soins infirmiers à domicile avec le financement de 4000 nouvelles places qui nous mettent sur la trajectoire d'augmentation de 20 % dont nous avons besoin d'ici à 2030 pour mieux les financer, nous proposons également d'adapter leur tarification pour mieux prendre en compte le profil des personnes accompagnées ensuite en renforçant la lisibilité de l'offre pour les Français en 2022 nous avons initié une logique de guichet unique en regroupant les différents services en 2023, nous vous proposons d'accélérer en incitant financièrement les services à dispenser à la fois des activités d'aide et de soins avec le forfait coordination développer le domicile, c'est aussi permettre aux professionnels de passer plus de temps auprès des personnes qu'ils accompagnent trop souvent, les intervenants ont tout juste le temps de faire les gestes élémentaires pour assurer le lever, le coucher, le repas est trop souvent les personnes qui les accueille ces interventions comme des temps mécanique minuté et déshumanisé, nous avons ouvert la discussion avec les départements pour pouvoir ajouter deux heures de présence supplémentaire chaque semaine auprès des 780000 personnes qui bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile. 2 heures dédiées à la convivialité et à la prévention 2 heures qui permettront aussi d'améliorer les conditions de travail des professionnels qui, trop souvent subissent des temps partiels ou du travail fractionné dans la continuité des travaux engagés à l'Assemblée nationale, le gouvernement présentera par ailleurs un amendement visant à introduire davantage de souplesse pour les bénéficiaires de la pas pour leur permettre de mobiliser davantage d'intervention à domicile. Développer le domicile, c'est enfin faire en sorte que l'inflation ne pèse pas sur le reste à charge de bénéficiaires l'année dernière nous avions instauré un tarif plancher à 22 euros de l'heure cette année nous faisons non seulement le choix de l'augmenter à 23 euros pour 2023, mais aussi de l'indexer sur la majoration tierce personne pour les années suivantes, c'est-à-dire sur un indice proche de l'inflation. Ces mesures permettent de diversifier l'offre de service sur nos territoire c'est également le sens de la priorité donnée au développement de l'habitat inclusif et à toutes les formes alternatives et innovantes qui permettent de s'adapter au parcours de vie des personnes, toutes ces mesures, nous les bâtissons avec les structures et avec leurs financeurs en 1er lieu les départements avec l'Assemblée des départements de France, nous avons réuni la semaine dernière un comité des financeurs, qui se réunira à niveau ce soir, nous y discutons de la mesure des deux heures dont j'ai déjà parlé et nous y aborderont notamment le soutien aux conditions de travail des aides, les services d'aide à domicile via notamment les concours de la CNSA aux conseils départementaux qui mérite d'être réformé. En ce qui concerne les moyens que nous consacrons aux personnes en situation de handicap, le gouvernement fait le choix d'une augmentation sans précédent : plus de 5,2 % c'est à la hauteur des ambitions que nous portons avec ma collègue Geneviève Darrieussecq pour tenir les engagements pris lors de la dernière conférence nationale du handicap et préparer la prochaine, qui se tiendra au tout début de l'année 2023 nous amplifions notamment la mise en oeuvre de grands objectifs pour l'école inclusive et la scolarisation des enfants et adolescents en situation de handicap pour l'accompagnement des adultes en situation de polyhandicap et des personnes handicapées vieillissantes et enfin, avec 80 millions d'euros supplémentaires pour des mesures concernant l'autisme et les troubles du neuro-développement nous prévoyons ainsi d'étendre aux 7 12 ans la politique de détection précoce qui est l'une des réussites majeures de la stratégie nationale et qui a permis à près de 30000 enfants depuis 3 ans, d'être détecté à temps et donc d'être correctement accompagné. Cet investissement prioritaire dans l'enfance se retrouve également dans la branche famille, pour laquelle nous proposons une augmentation exceptionnelle d'un milliard 600 millions d'euros, c'est un choix fort du gouvernement, qui rejoint 2 objectifs au coeur du projet du président de la République, le plein emploi et l'égalité des chances, pas de plein emploi dans une société où trop souvent des femmes doivent renoncer à travailler faute de modes d'accueil adaptés pour leurs enfants, pas d'égalité des chances non plus dans une société qui reproduit les inégalités en ne soutenant pas les familles les plus fragiles, concrètement, nous proposons de réformer l'aide à la garde individuelle d'enfant le complément mode de garde dans les familles, ils connaissent bien l'importance en faisant 2 choses : d'une part en modifiant le barème pour permettre aux familles qui ne recourt pas à la crèche, de pouvoir faire garder leur enfant au même coût par une assistante maternelle ou une garde à domicile en emplois Directs. Et d'autre part, en rallongeant son bénéfice au-delà de 6 ans et jusqu'à l'entrée au collège pour les familles monoparentales, c'est un choix fort que nous assumons d'apporter une attention toute particulière aux familles monoparentales, dont 30 % vivent dans la pauvreté et 90 % sont des femmes. C'est ce même engagement aux côtés des familles monoparentales qui nous a conduit à augmenter, il y a quelques jours, de 50 pour 100 la pension alimentaire minimale de 123 à 185 euros par mois et par enfant. Voilà Mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs, les grandes mesures de ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale, ces mesures vont changer concrètement la vie de millions de femmes et d'hommes, elles vont permettre de soutenir des professionnels éprouvés par la crise et que nous devons accompagner dans les grandes transformations elle contribue aux réformes structurelles du quinquennat pour que notre modèle social répondent mieux aux besoins des Français, c'est le cas de mesures famille qui s'inscrivent dans la droite ligne de la politique des 1000 premiers jours et qui sont une brique de service public de la petite enfance, cette grande réforme, nous allons la construire avec les collectivités locales tout au long du quinquennat pour que chaque famille puisse avoir une solution d'accueil de qualité pour ses enfants, c'est aussi le cas des mesures autonomie qui s'inscrivent dans le chantier plus global que nous avons ouvert pour préparer la société dans toutes ses dimensions au vieillissement de la population, j'étais vendredi dernier à Châlons en Champagne pour animer le premier atelier territoriale du Conseil national de la refondation dédié au bien-vieillir autour de cette question si fondamentale, l'une des plus cruciales à laquelle nous devons répondre dans les prochaines années, nous avons réuni des élus, des professionnels de tous les secteurs, des personnes âgées et leur famille, c'est des acteurs associatifs et privés pour construire des solutions opérationnelles directement sur les territoires. C'est ce même esprit de pragmatisme et d'ambition que porte ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale, c'est cette même méthode d'écoute et de co-construction que je vous propose, pour en discuter ensemble, je vous remercie. Merci, monsieur le Ministre. La parole est maintenant madame Olivia Grégoire Ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, vous avez la parole madame la Ministre. Merci monsieur. Monsieur le président, madame la présidente, madame la rapporteure générale. Madame messieurs les Ministres, mesdames, messieurs les sénateurs, au nom de mes collègues du gouvernement et du ministre Gabriel Attal dont je vous prie de bien vouloir excuser l'absence puisqu'il est retenu comme vous le savez, à l'Assemblée nationale pour l'examen actuellement du second projet de loi de financement rectificative pour 2022, permettez-moi d'exprimer on une journée un peu particulière pour moi au plan personnel, j'ai l'honneur d'être la fille d'un papa qui a été très lourdement accidenté en 7 novembre 1985. Je n'aurais Guillermo je sais dans ma chère, ce que nous devons à nos professionnels de santé. Et au-delà de la considération que nous avons toutes et tous pour eux, on a eu l'occasion de voir dans les épisodes extrêmement douloureux du Covid à quel point leur présence, leur engagement et tête absolument irréprochable. évidemment, l'État a été présent, il a répondu présent, vous le savez, tout aussi bien que moi, mesdames, messieurs les sénateurs, au travers du quoi qu'il en coûte, il a évité à notre pays un cortège de difficultés, c'est ensemble que nous avons pu traverser cette épreuve très difficile de la pandémie, bousculé par le choc, notre société a aussi su trouver les ressources, les ressorts pour résister la responsabilité qui nous incombe désormais. C'est de poursuivre la reconstruction, comme l'a dit à l'instant le ministre Brown, il nous faut bâtir ensemble un un système plus solide, plus accessible, plus efficace, plus juste, plus accessible, c'est d'abord et avant tout améliorer l'accès aux soins, l'effort ne débute pas aujourd'hui depuis 2017 les forces chiffre nous avons investi 53 milliards d'euros de plus dans notre système de santé avec un Ondam, passer de 191 milliards d'euros en 2017 à 244 milliards d'euros en 2023, nous avons mis fin aux baisses de tarifs hospitaliers nous avons déployé le 100 % santé supprimer le numerus clausus soutenu l'aide à domicile et n'osaient pas des nous allons poursuivre cet effort, conformément aux engagements qui ont été pris devant les Français, c'est pourquoi, avec ce Plfss l'Ondam progressera en 2023 à un niveau historique de 3 7 % une progression de 50 % plus rapide qu'au cours de la décennie 2010 pour l'Ondam hospitalier, l'augmentation sera de 4 virgule un pour 100 en 2023, c'est 2 fois plus qu'au cours de la décennie 2010, elle finance notamment, vous le savez, une enveloppe exceptionnelle de 800 millions d'euros en 2000 22 et 800 millions d'euros supplémentaires en 2023 concertée par mon collègue François Braun avec les fédérations hospitalières et médico- social en ville, nous encouragerons le cumul emploi-retraite des médecins proches de la retraite ou en retraite, comme durant la crise sanitaire, cette incitation prendra la forme d'une exonération de cotisations vieillesse pour 2023, dans l'attente des conclusions du CNR santé renforcer l'accès aux soins, c'est aussi mieux prendre en charge nos aînés indépendants comme vient de le rappeler, le ministre Combe avec un Ondam médico-social à plus 5 1 % en 2023, nous finançons le plein effet des augmentations de salaire, l'embauche de milliers de soignants et l'investissement pour les services à domicile, je rappelle que les augmentations salariales qui ont été décidées depuis la crise sanitaire, représente un effort de 3,2 milliards d'euros par an pour la 5ème, branche que nous avons créée en 2021, nous agissons pour faciliter l'accès aux modes de garde parce que nous savons combien le destin de nos jeunes enfants se joue des leurs 1000 premiers jours ce PLFSS il pose la première Pierre d'un véritable service public de la petite enfance, en réduisant drastiquement le reste à charge des familles pour le recours aux assistants maternels, très concrètement, un couple de classe moyenne qui confie son enfant 50 heures par semaine économisera quasiment 2000 euros sur une année, c'est du pouvoir d'achat pour des dizaines de milliers de familles et cela s'ajoutera à la hausse du plafond du crédit d'impôt, garde d'enfants, que vos collègues députés ont relevé de 2003 à 3500 euros en PLF 2023, tous ces progrès, mesdames, messieurs les sénateurs ne sont possibles, vous le savez, que si nous continuons à donner la priorité au travail et à la production, les cotisations, socle du financement de l'Sécurité sociale vont progresser de 391 milliards d'euros en 2022 à 407 milliards d'euros en 2023 et nous le devons aux créations d'emplois, 310000 sont prévues en 2022 220000 déjà réalisées au seul 1er semestre 117000 supplémentaires attendus en 2023 au total de 2020 à 2023 malgré la crise, notre pays pourrait créer 1,2 millions d'emplois n'oublions jamais, et je sais que vous ne l'oubliez pas que c'est le travail qui tient le financement de notre système social, voilà pourquoi ce PLFSS entend rendre notre système social plus efficace parce que les besoins sont immenses, on ne doit ménager aucun effort pour trouver des marges d'efficience, hé oui pour réaliser aussi des économies là où elles sont pertinentes et elles peuvent être substantielles, gouverner c'est choisir, vous le savez c'est pourquoi nous assumons de demander des efforts à certains acteurs qui peuvent contribuer à l'effort commun nous assumons de demander des efforts aux laboratoires de biologie qui ont réalisé cette 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires au titre des tests Covid en 2020 et 21 et nous saluons évidemment leur mobilisation sans faille durant la crise, ils bénéficiaient avant crise d'une rentabilité très élevée de près de 30 % et la CNAM négocie INRA une baisse de prix avec le secteur pour au moins 250 millions d'euros dès 2023, nous assumons aussi de demander des efforts à l'imagerie médicale, qui représente près de 5 milliards d'euros de dépenses où nous pouvons limiter les examens redondants inapproprié ou parfois inutile, nous demanderons à la CNAM de négocier là aussi un nouveau protocole pour juguler la dépense de 150 millions d'euros en 2023, nous assumons enfin de demander des efforts aux fabricants de médicaments, les dépenses de médicaments sont dynamiques, le fait du vieillissement démographique et de l'arrivée aussi de nouvelles molécules sur le marché, c'est de s'il signe que nous devons redoubler d'efforts pour la pertinence des prescriptions et les baisses de prix ciblé sur les médicaments les plus anciens pour dans le même temps mieux récompenser l'innovation ces baisses de prix s'élèveront à 800 millions d'euros en 2023 ces efforts, nous ne les demandons pas par plaisir de faire des économies, nous les demandons parce qu'ils sont indispensables pour dégager des marges de manoeuvre budgétaires et justement mieux investir dans l'hôpital, en ville comme dans le médico-social, soyons très clair, quand nous parlons d'économie, il s'agit d'effort de maîtrise par rapport à des dépenses qui continueront d'augmenter, ils sont la condition pour garantir la soutenabilité la résilience de nos comptes sociaux, je rappelle que les taux d'intérêt à 10 ans pour ceux qui l'oublieraient les taux d'intérêt à 10 ans sur la dette française frôle les 3 % ceux du Royaume-Uni dépasse les 4 % et ceux de l'Italie se rapproche des 5 la parenthèse de l'argent gratuit sur les marchés, c'est bel et bien refermée, retrouver une trajectoire maîtriser de nos comptes publics et la condition sine qua non de notre indépendance financière enfin et pour terminer, mesdames, messieurs les sénateurs, nous voulons avec ce Plfss construire un un système qui soit plus juste assurer la justice est aussi adressé un message de fermeté à l'égard de tous les fraudeurs et je sais qu'en tant que sénatrice et sénateurs, vous y êtes attachés depuis longtemps, qu'il s'agisse d'ailleurs de la fraude aux cotisations ou aux prestations puisque les fraudes se perfectionne, nous allons aussi nous perfectionner nous allons perfectionner les outils de notre lutte avec des pouvoirs de Cyber enquête confiée à plus de 400 contrôleurs des caisses de Sécurité sociale pour mieux repérer et réprimer les fraudes à enjeu avec les échanges d'informations qui vont être renforcées, notamment entre les greffiers des tribunaux de commerce et les caisses de Sécurité sociale et en reprenant aussi une proposition émise par votre chambre, nous interdirons le versement de prestations sociales, hors pensions sur des comptes bancaires qui ne seraient pas situés en zone c'est pas puisque ces prestations sont soumises à condition de résidence sur notre territoire, je sais que ce sujet a fait l'objet d'un rapport de votre commission des affaires sociales, je veux vous en remercier le texte qui vous est soumis propose justement des dispositions sur le transfert Agirc Arcco je veux à cet égard rappeler rapidement que le texte qui vous est soumis répond précisément à la recommandation des sénateurs formulées dans le rapport que je viens de citer ça varie à pour Sow puisque nous reportons à 2024 le transfert du recouvrement des cotisations de retraite complémentaire aux Urssaf, c'était aussi la demande des syndicats et du patronat, deuxièmement nous demandons à l'Agirc-Arrco et aux Urssaf de conclure une convention pour inscrire leur partage de responsabilités, noir sur blanc, je vais être très clair, le métier des Urssaf et de recouvrer des cotisations, pas de verser des retraites ni aujourd'hui ni demain les Urssaf ne verseront les retraites complémentaires, l'Agirc Arcco continuera à fiabiliser les données personnelles des salariés, enfin ce transfert s'inscrit dans le mouvement d'unification du recouvrement social au sein du Urssaf et du recouvrement fiscal à la DGFIP, c'est l'une démarche de simplification des entre, pour les entreprises, avec un objectif de gain de recouvrement pour le régime Agirc Arcco lui-même, mesdames, messieurs les sénateurs, au cours de nos débats, je n'en doute pas, nous allons enrichir ensemble ce PLFSS et sur ces bancs, je crois que vous partagez l'objectif de refondation et de consolidation de notre système social d'entre vous et force de proposition sur ces enjeux, vous l'avez démontré et, au-delà de nos clivages légitime, sachons bâtir avec confiance, mais aussi responsabilité un Plfss qui soit une brique importante d'un système social plus efficace, plus juste et plus solidaire, je vous remercie. Merci madame la ministre, La parole est maintenant Madame Agnès Firmin Le Bodo Ministre délégué chargé de l'organisation territoriale et des professions de santé. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, madame la présidente de la commission madame la rapporteure, mesdames et messieurs, le les sénateurs, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, c'est l'effort collectif consacré par notre nation pour protéger la collectivité face aux aléas de la vie, aux côtés de mes collègues, la ministre en charge de l'organisation territoriale et des professions de santé que je suis être honoré de présenter aux spécialistes des territoires que vous êtes des engagements forts de ce PLFSS. Alors que notre système de santé a été fortement sollicitée et qu'il a su relever le défi de la crise sanitaire grâce à l'engagement sans faille de l'ensemble des acteurs de santé que je tiens, ici, une nouvelle fois à saluer ce PLFSS porte une ligne claire celle de la défense des préoccupations essentielles de nos concitoyens plus de prévention, un accès renforcé aux soins, un système plus juste et plus éthique ce PLFSS porte ainsi des mesures fortes en matière de prévention avec le nouveau rendez-vous aux âges clés de la vie ou pour améliorer la santé des femmes de dépenses de défense de l'hôpital très éprouvés par la pandémie et qui a porté à bout de bras par tous les personnels soignants le PLFSS le ministre François Braun a longuement évoqué le gouvernement a pris ses responsabilités en reprenant une partie de la dette hospitalière pour redonner de l'air aux établissements et leur permettre d'investir les engagements inédit du Ségur de la santé ont apporté une réponse forte à la demande légitime de reconnaissance et de valorisation de l'engagement des soignants, ces efforts se prolonge dans ce PLFSS nous leur donnons aussi de nouveaux outils pour encadrer l'intérim qui fragilise les équipes et pèse sur les comptes des hôpitaux, nous avons également pris à bras le corps la question de l'intégration des personnels de santé étrangers, c'est une priorité de mon ministère par amendement à l'Assemblée nationale, le gouvernement a souhaité déclarer dès que l'aller au 30 avril prochain la date butoir de régularisation des pas du soumis au Cadre les cales de la loi de santé de la pandémie a porté, vous le savez, un coup d'un coup d'arrêt au processus d'évaluation et de reconnaissance de leurs compétences en responsabilité cette date limite avait été reporté une première fois au 31 décembre 2022, notre objectif, ce n'est pas de pénaliser les hôpitaux et les patients au sein desquels ces praticiens jouent souvent un rôle essentiel dans la continuité des soins, c'est aussi de conserver toutes les exigences nécessaires sur le niveau de compétence requis, c'est garder toujours à l'esprit que les femmes et les hommes que l'on appelle les pas du participe pleinement au fonctionnement de notre système de santé, c'est enfin un PLFSS qui traduit notre engagement en matière d'accès aux soins et de lutte contre les déserts médicaux à travers une simplification des aides à l'installation via le guichet unique de nouvelles mesures pour favoriser le maintien en activité des médecins et encore l'introduction de la notion de responsabilité collective en matière de permanence des soins. nous notre modèle de protection sociale c'est aussi agir avec responsabilité contre toutes les formes de fraude comme vient de l'évoquer ma collègue Olivia Grégoire la fraude, je le dis nettement, c'est un coup bas porté à notre pacte républicain et à la justice sociale, parce qu'elle sape le consentement à l'impôt, elle pénalise en priorité, les Français les plus modestes, c'est-à-dire tous ceux qui bénéficient légitimement de nos filets de sécurité lutter contre les fraudes, c'est aussi une exigence forte pour garantir la pérennité de notre modèle, avec mon collègue Gabriel Attal, nous avons souhaité porter plusieurs mesures dans ce PLFSS en s'appuyant sur de nouveaux outils, il s'agit à la fois de mieux prévenir et détecter les fraudes, je pense à l'élargissement des possibilités de déconventionnement d'urgence des professionnels de santé, en cas de violation grave des engagements conventionnels ou à la mise en place d'un nouveau barème de pénalités financières en cas de fraude à cet égard, l'article 44 du PLFSS sur l'extrapolation a peut-être été mal compris, il s'agit en effet d'une mesure qui vise avant tout à chiffrer au plus près le préjudice de l'assurance maladie qui ne peut aujourd'hui contrôler qu'une fraction limitée des factures, cette mesure avait étant proposée par la Cour des comptes en 2020. Parce que ce PLFSS est ambitieux : je me réjouis de l'ouverture de ces débats devant votre assemblée, je sais le Sénat attentif à l'équilibre des comptes sociaux, condition essentielle à la pérennité de notre modèle je vous sais aussi particulièrement attaché à la prise en compte des réalités des territoires ce PLFSS est une première étape qui sera complété par le CNR en santé qui se déploient en ce moment sur l'ensemble du territoire en poursuivant l'objectif non seulement de mettre en valeur toutes les initiatives locales déjà existantes, mais également de trouver des solutions nouvelles pour notre système de santé, je vous remercie. Merci madame la ministre. La. Parole est maintenant à Madame Élisabeth Doineau, rapporteur général de la commission des affaires sociales pour dix minutes. Merci monsieur le président, Mesdames, messieurs les Ministres, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur pour avis de la commission des finances, mes chers collègues, nous nous apprêtons à examiner 1er projet de loi de financement de la Sécurité sociale de la législature, ces conditions d'examen par l'Assemblée nationale ont été particulières, vous n'allez pas me contredire, les députés ont tout d'abord rejeté les 1ère et 2ème partie du texte relative au compte du dernier exercice clos et à la rectification des prévisions de recettes et aux objectifs de dépenses de l'année en cours 2022, par la suite, le gouvernement a engagé à 2 reprises sa responsabilité, en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, une première fois sur la 3ème partie du texte relative aux recettes de l'année à venir avant même d'avoir commencé l'examen de cette partie une seconde fois sur la quatrième partie relative aux dépenses de l'année et à venir sur l'ensemble du PLFSS après avoir examiné quelques articles concernant pour l'essentiel, la branche autonomie, il en résulte que le Plfss pour 2023 nous arrive tronqué vidé de ses 2 premières parties, ce qui est assez inédit que le gouvernement n'a pas pu rétablir quand il a engagé sa responsabilité sur les parties suivantes surtout le débat parlementaire lui-même a jusqu'à présent été tronqué au vu des enjeux financiers et politiques particulièrement important des projets de loi de financement de la Sécurité sociale, nous avons donc la responsabilité de faire vivre au Sénat des débats complet sur le PLFSS pour 2023, soyez sûrs, mesdames, messieurs les ministres, que ce débat seront à l'image du Sénat c'est-à-dire sérieux et respectueux mais aussi exigeant et parfois en contradiction avec votre approche, j'en arrive au compte-tenu de ce projet de financement de la Sécurité sociale, comme l'ont dit les ministres, les comptes de la Sécurité Sociale s'améliore depuis le trou d'air historique de l'année 2020, pic de la crise sanitaire, économique et sociale provoquée par l'épidémie de Covid 19 de ce point de vue, le gouvernement considère que l'année à venir 2023 devrait de nouveau marqué une progression avec un déficit réduit à 7,2 milliards d'euros, cela reste significatif, bien sûr, pour des comptes censé être équilibré, mais nous sommes loin des quelque 39 8 milliards d'euros de 2020 record historique de déficit des comptes sociaux nous en acceptons l'augure cependant notre commission a exprimé son inquiétude face aux chiffres que vous nous présentez inquiétude quant à la crédibilité des comptes pour 2023 tout d'abord le tableau d'équilibre repose sur des hypothèses que le Haut Conseil des finances publiques, qualifie d'optimiste d'une part pour ce qui concerne les recettes, le gouvernement prévoit une croissance du PIB de 1 % et une nouvelle progression de la masse salariale à 5 d'autre part pour ce qui concerne les dépenses, le gouvernement prévoit une quasi-disparition des dépenses liées au Covid 19 la provision correspondant à seulement 1 milliard d'euros, ça nous semble un peu faible, ce qui devrait là aussi être vérifié et nous comptons nous donner les moyens de le faire et nous comptons vous donner les moyens de le faire, vous ne comptait d'ailleurs que sur cette vision optimiste de la conjoncture économique et sanitaire pour tenir les comptes et pas sur les mesures que vous prendrez à cet égard, il est significatif que le solde que nous transmet l'Assemblée nationale est égal au solde tendanciel, c'est-à-dire au sol de que l'on constaterait sans prendre aucune mesure en définitive au niveau de ce Plfss notre inquiétude aussi pour l'avenir, en effet, si l'on se penche au-delà de 2023, au travers de ce que propose l'annexe B qui quadriennal de ce Plfss, on peut observer que le déficit relativement modeste espérer pour 2023 ne devrait être qu'une étape sur le chemin du retour à l'équilibre, mais bien plutôt une simple embellie avant un nouveau creusement des déficits, selon vos propres prévisions, la situation des comptes de la Sécurité Sociale devrait se dégrader dès 2000 24 à un niveau de de moins 8 8 milliards d'euros mais surtout atteindre un niveau plus tard plus inquiétant autour de 12 milliards d'euros de déficit par an 2020 en 2025 et 2026 or tout ce scénario repose là aussi sur des hypothèses de croissance optimistes et des perspectives de maîtrise des dépenses, notamment sur l'Ondam dont nous ne savons rien ainsi l'annexe B qui a aussi pour vocation de donner une visibilité et une stratégie pour l'avenir ne donne aucun détail sur les moyens que le gouvernement envisage de se donner pour maîtriser les comptes par exemple, il est tout juste préciser que le solde de la branche vieillesse, bénéficieraient de l'objectif d'élévation progressive de l'âge effectif de départ sur le quinquennat le Haut Conseil des finances publiques, déplore lui aussi que vos prévisions supposent des effets importants et immédiats de réformes dont ni les modalités ni les impacts, ni le calendrier ne sont documentés, en somme, cette trajectoire qui devrait se dégrader dès 2000 vingt-quatre reste hélas une version optimiste de l'avenir des comptes sociaux, il est donc à craindre que les déficits continuent de s'accumuler et que de nouveaux transferts la s'doivent être envisagées à l'avenir dans cette situation, la commission des affaires sociales a adopté une approche responsable de ce Plfss pour la résumer en quelques mots : la commission proposera tout d'abord, de rétablir les parties de loi de financement de la Sécurité sociale, qui doivent exister, quitte à les corriger, comme en première partie de marquer notre refus de la vision que le gouvernement présente de l'avenir de la sécurité sociale à l'annexe B à la sincérité douteuse et à la dimension stratégique absente de poser nous-mêmes des jalons de véritables mesures d'équilibre en particulier sur les retraites, mais aussi en proposant quelques recettes supplémentaires et de renforcer enfin le contrôle du Parlement, notamment dans le cas où les hypothèses optimistes du gouvernement ne se vérifierait pas par exemple en cas de dépassement significatif de l'Ondam et des dépenses d'urgence, vous l'aurez compris, mesdames, messieurs les Ministres, nous serons tout au long de ce débat que nous espérons riche des interlocuteurs à la fois exigeant mais constructif, et quelquefois c'est nécessaire si nécessaire des contradicteurs, je vous remercie de votre attention. Merci madame la rapporteure générale, la parole est maintenant Madame Corinne Imbert, rapporteure de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie. Pour cinq minutes. Vous avez la parole cher collègue.

Monsieur le président, mesdames les ministres, messieurs les Ministres, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure générale, mes chers collègues, ce budget de l'assurance maladie et le 3ème depuis le déclenchement de l'épidémie de Covid 19 et le 1er de la nouvelle équipe départ gouvernementale pardon je pas rabaisser le gouvernement au département, monsieur le Ministre, vous imaginez bien la la première circonstances pourrait commander une certaine prudence dans le cadrage financier, la seconde un peu d'audace dans les mesures nouvelles, hélas, nous n'avons trouvé ni l'une ni l'autre, la trajectoire financière d'abord est improbable, le redressement annoncé à spectaculaire mais il résulte d'un effet recettes anticipées sur la base non pas de mesures nouvelles mais d'hypothèses tant macro-économique qui épidémiologique très optimiste, la dépense dans le Champ de l'Ondam seraient en baisse en tenant compte des dépenses Covid mais elle augmenterait de 3 7 % hors Covid selon un rythme de progression soutenue dans tous les sous-objectifs 2 9 % pour les soins de ville 4 virgule un pour 100 pour les établissements de santé, notamment derrière ces dynamique de dépenses, pourtant, on peine à distinguer une grande politique de soutien au système de santé l'Ondam hospitalier par exemple n'est porté que par la revalorisation du point d'indice et la forte inflation dans 5 ans, l'Ondam atteindrait ainsi 270 milliards d'euros, alors qu'il dépassait à peine les 200 milliards en 2019, progressant de plus de 6,5 milliards d'euros par an, c'est impressionnant, mais à quoi correspondent ces montants, ce ne sont pas les professionnels de santé, ni ceux qui cherchent à les consulter, qui saurait le dire la crédibilité de ce budget est ainsi mise en cause et je n'ai même rien dit de la sincérité de la discussion parlementaire lorsque de jeunes héros annonce médiatique interviennent en plein examen les mesures nouvelles, non par ailleurs par le niveau d'ambition qu'exige notre système sanitaire, voyez la prévention, l'article 17 est à lui seul, ou presque, l'emblème d'une nouvelle intitulé du ministère, rebaptisé de la santé et de la prévention, or il est peint en trompe oeil puisque des 3 rendez-vous de prévention tout au long de la vie à 20 à 25 40 45 et 60 65 ans que promet le dossier de presse, le 3ème est déjà en cours de déploiement et le deuxième ne prendra la forme que de rendez vous ou de séances assez indéterminé, la prévention est une chose trop sérieuse et dans notre pays, trop urgente pour creuser à ce point l'écart des promesses aux réalisations en matière d'accès aux soins de ville, les mesures existent mais elles sont timides brouillonne, les 2 qualificatifs n'étant pas mutuellement exclusifs à l'heure où tout semble prêter le flanc le refondation l'article 22 prétend plus modestement rénover la vie conventionnelle, en réalité il ne modifie qu'à la marge les règles encadrant les conventions conclues entre les organisations représentatives des professions de santé et l'assurance maladie, le texte nous en doute parvenue bardé d'un certain nombre d'articles additionnels parfois à la limite de la recevabilité et composant davantage qu'une loi de financement, une espèce de loi santé en costume d'Arlequin, avec accès Direct aux infirmiers en pratique avancée, élargissement de la permanence des soins dépistage la drépanocytose expérimentation de consultations avancées certificat de décès tous ces sujets sont bien sûr importants mais il gagnerait à être examinées de manière cohérente à l'abri des contraintes pesant sur le calendrier budgétaire sur ces aspects, comme sur celui-là téléconsultation que le gouvernement propose de mieux encadrer, nous proposerons néanmoins des améliorations, ainsi que le rétablissement du dispositif de la proposition de loi du président Retailleau sur la quatrième année de médecine générale mais, curieusement, aucune mesure de cette loi de financement ne concerne le financement de l'hôpital, la seule mesure relative à l'hôpital, concerne l'interdiction de l'intérim médical, notamment pour les jeunes diplômés, médecins et infirmiers c'est souhaitable, mais l'intérim des jeunes diplômés, n'est pas le seul à fragiliser le fonctionnement des établissements de santé, la qualité et la continuité des soins, nous proposerons d'aller plus loin quant aux mesures de régulation des produits de santé, de la biologie médicale, elles étaient manifestement mal préparé, le gouvernement a ainsi finalement supprimer la contribution spécifique aux médicaments en forte croissance et rééquilibrer en contrepartie la clause de sauvegarde en plafonnant les contributions du pour l'année 2023, il a en outre abandonné le référencement périodique des médicaments que les fabricants et pharmaciens avaient jugé dangereux et inadapté. L'article 27, lui, s'apparente à rien moins qu'y a une une un ultimatum, c'est au secteur de la biologie médicale puisque, à défaut d'accord, un arrêté ministériel fixerait une baisse généralisée de la cotation des actes une contribution exceptionnelle assise sur le remboursement du dépistage du Covid en 2021 nous semble plus juste, vous le voyez, mes chers collègues, la déception est grande, sous réserve du vote des modifications issues des travaux de la commission je vous proposerai sans grand enthousiasme, comme je l'ai dit, dans la commission d'adopter ce projet de loi de financement dans son volet assurance-maladie je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est maintenant à la présidente, Pascale Gruny, rapporteur de la commission des affaires sociales pour les accidents du travail et les maladies professionnelles pour cinq minutes.

Monsieur le président, Mesdames et messieurs les ministres, madame la présidente, madame la rapporteure générale, Madame et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues excédentaire depuis 2013, la branche accidents du travail-maladies professionnelles AT-MP a renouer avec cette situation en 2021 après une année de déficit exceptionnel ce rebond se confirme en 2022 pour 2023, l'objectif de dépense de la branche AT-MP est fixé à 14 8 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base le PLFSS confirme le retour à une situation financière favorable avec un excédent de 2 2 milliards d'euros à moyen terme, l'écart entre les recettes et les dépenses s'amplifierait atteignant 3,3 milliards d'euros en 2026 cette situation qui peut sembler confortable signifie surtout que le calibrage des recettes de la branche AT-MP reste structurellement déconnecté de ses besoins de financement, le ratio d'adéquation des recettes aux dépenses dépasseraient 120 % en 2026 en l'absence de mesures nouvelles, des mesures de rééquilibrage doivent donc être envisagées, elles peuvent passer par de nouvelles dépenses, notamment en matière de prévention et par la poursuite de l'ajustement à la baisse des cotisations, il me semble important de réaffirmer, mesdames et messieurs les Ministres, que les excédents de la branche ne doivent pas être utilisée pour d'autres finalités que la prévention et et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, malgré ses marges financières le PLFSS ne contient cette année que peu de mesures affectant signifie significativement de dépenses, il améliore la couverture des non-salariés agricoles pluriactifs en leur permettant de promo de percevoir des indemnités journalières maladie au titre de l'activité non salariée qui ne peuvent pas exercer en cas d'accident ou maladie professionnelle dans le cadre d'une activité salariée, en sus des indemnités journalières AT-MP dont il bénéficie à ce titre en outre cet article permet aux conjoints collaborateurs et aux aides familiaux de bénéficier d'une rente AT-MP en Cada capacité permanent partiel ces mesures à l'impact financier très limités sont néanmoins bienvenue par ailleurs 2 articles additionnels ont été retenues par le gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, il procède à des ajustements très ponctuel du dispositif d'indemnisation par le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides des enfants atteints d'une pathologie causée par leur Exposition prénatale du fait de l'activité, l'activité professionnelle de leurs parents, cette indemnisation reste marginal dans l'activité du fonds créé en 2020 est adossée à la MSA cette demande déposée en 2021 et seulement de suite favorable de manière classique, le PLFSS fixe les montants des transferts versements de la branche AT-MP au Fonds amiante et vers d'autres branches, le montant du versement de la branche maladie au titre de la sous-déclaration des AT-MP serait fixé à 1 virgule 2 milliards d'euros pour 2023 alors qu'il était de 1,1 milliard d'euros en 2022, et d'un milliard d'euros les 7 années précédentes cette augmente, hein, cette augmentation de temps annoncé l'an dernier par le gouvernement vise à approcher le point bas de l'estimation de la commission chargée d'en évaluer tous les 3 ans, le coût réel pour la branche maladie, or le nombre de maladies professionnelles a diminué de plus de 10 % entre 2012 et 2021, des progrès ont été accomplis en matière de sensibilisation, d'information apportée aux victimes et de simplification des procédures dans ce contexte, l'augmentation de ce versement apparaît comme une ponction réalisée dans des conditions peu transparente qui ne vise qu'à contribuer à combler le déficit de la branche maladie, imagine-t-on qu'une autre caisse soit tenus de payer le coût supposé du non-recours aux prestations qu'elle est chargée de verser la commission propose donc, comme l'an passé, de réduire le montant de ce versement à un milliard d'euros, ce qui nous semble représenter un maximum les 200 millions d'euros ainsi conservé par la branche pourrait utilement être fléché vers la prévention et l'accompagnement quant au montant des dotations au Fonds amiante : le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et le Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, il augmente en valeur absolue de 547 à 557 millions d'euros, mais son poids relatif dans l'ensemble des dépenses de la branche continue continue de décroître en cohérence avec la baisse tendancielle du nombre des travailleurs ayant été exposés à l'amiante au cours de leur carrière sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle a déposé la commission vous invite à approuver l'objectif de dépense de la branche fixé à 14 8 milliards d'euros pour 2023 je vous remercie. Merci madame la présidente remarquables. La parole est maintenant Monsieur René-Paul Savary, rapporteur de la commission des affaires sociales pour l'assurance vieillesse pour cinq minutes. Merci, cher collègue. Année après année, l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale et l'occasion pour le Sénat d'alerter le gouvernement à propos de la dégradation de la situation financière de la branche vieillesse année après année, nous assumons nos responsabilités et adoptons les mesures difficiles que les circonstances imposent pour garantir le versement des pensions dans la durée et éviter à nos enfants d'avoir à travailler au-delà de 65 ans, année après année, le gouvernement se voile la face en reportant sans cesse où l'on demain l'une des décisions les plus importantes qu'il est à prendre, il y a 5 ans, souvenez-vous, le candidat Emmanuel Macron estimait qu'il n'y avait pas de problème de financement du système de retraite. Le temps a passé, les déficits se sont accumulés et un beau jour, telle la vigie du Titanic, le président de la République a finit par apercevoir les icebergs, c'est à nous désormais qu'il revient de fermer en urgence les cloisons étanches pour maintenir la France à flot, en effet, la situation de la branche vieillesse n'autorise plus la moindre tergiversations, le vieillissement démographique, le ralentissement de la croissance, la persistance d'une inflation soutenue devrait porter son déficit à 13 6 milliards d'euros d'ici 2026, notons que cette projection intègre les effets d'une réforme des retraites dont le gouvernement n'a pas daigné me communiquer les paramètres exacts et dont on sait uniquement qu'elle améliorer le solde de la branche de 8 à 9 milliards d'ici 2027 face à un horizon aussi chargé le PLFSS 2023 ne contient quasiment aucune mesure ayant une incidence financière sur la branche, hormis quelques articles portant sur la lutte contre la fraude sociale qui ne générerait que quelques millions d'euros de recettes supplémentaires au profit de la branche, dans ce contexte, je proposerais à notre assemblée d'instituer une convention nationale pour l'emploi des seniors et la sauvegarde du système de retraite. Rassemblant des représentants des partenaires sociaux de l'État, des associations familiales de retraités ainsi que des personnalités qualifiées, cette instance sera chargée de proposer au gouvernement des mesures tendant notamment à favoriser le maintien des seniors dans l'emploi, un oeil nouveau une vision nouvelle des seniors dans notre société, garantir la prise en compte de la pénibilité du travail, du handicap des carrières longues dans leur définition et ramener la branche vieillesse à l'équilibre à l'horizon 2033 vivement aboutissait à un compromis sur des mesures permettant d'atteindre ses objectifs, un projet de loi les incluant devrait être proposé sans délai devant le Parlement en cas d'échec des discussions, ce que ne regrette rien, plusieurs mesures paramétrique entrera en vigueur le 1er janvier 2024, il s'agirait ainsi de fixer dans la loi l'âge du taux plein automatique à son niveau actuel, soit 67 ans, il est pas inscrit actuellement dans la loi de porter la durée de cotisation à 43 unités dès la génération 1967 au lieu de la génération 1973 ce qui représenterait près de 3 milliards d'euros de recettes supplémentaires à l'échec du système de retraites à l'horizon 2030, de reporter de 2 ans l'âge légal de départ pour atteinte 64 ans, 64 à compter de la génération 1967 ce qui améliorerait le solde de système de retraite toujours à l'horizon 2030, de près de 13 milliards d'euros. Bien entendu, cette réforme concernerait également les régimes spéciaux qui devront contribuer autant que les autres à l'effort collectif et ce, bien sûr, avant 2033 je vois dans ces mesures, le seul moyen de ramener la branche vieillesse à l'équilibre, sans augmenter les cotisations, ni diminuer les pensions à défaut nous laisserions à la jeunesse, un système de retraites en bien piètre état avec, selon les estimations du comité d'orientation des retraites, un déficit de de 45 milliards d'euros en 2070 nous rendrons-nous coupables d'une telle négligence et j'ose le dire, d'une telle lâcheté, je ne peux pas le croire alors, mes chers collègues, laissons de côté les clivages partisans et unissons-nous autour de ce qui nous rassemble souvent ensemble notre système de retraite, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est maintenant monsieur Olivier Henno, rapporteur de la commission des affaires sociales pour la famille, pour cinq minutes.

pour l'exercice 2022, la branche famille sur un excédent de 2,6 milliards d'euros, il se réduirait de moitié en 2023 pour atteindre 1,3 milliards d'euros cet amoindrissement de l'excédent résulte pour 850 millions d'euros de la décision bienvenue du gouvernement de revaloriser de moitié l'allocation de soutien familial en faveur des parents isolés, c'est l'une des rares lueurs de ce Plfss pour les 70 % restants la baisse provient du transfert, la CNAF de la charge des indemnités journalières du congé post-natal de maternité cette mesure grève les dépenses de 2 milliards d'euros, sans que les familles n'y trouve concrètement le moindre Avantage la trajectoire financière plus annuel de la branche en serait fortement affectée avec un excellent réduit à 500 millions de 1000 25, privant la branche famille, des moyens d'une ambition nouvelle c'est pourquoi l'initiative de la rapporteure générale, la commission vous proposera de supprimer ce transfert de charges, cela dit, s'agissant des articles concernant la branche famille ce PLFSS concentre se concentre sur la réforme de complément de libre choix du mode de garde 10 CMG le CMG emplois Directs compense aux familles, le coût de la garde de leurs enfants, âgés de moins de 6 ans lorsqu'elle recours à une assistante maternelle ou à une personne salariée pour une garde à domicile, le barème actuel induit des effets de seuil important et provoque des restes à charge élevés pour les foyers aux revenus les plus modestes, il rend quasiment impossible le recours à un mode de garde individuel pour ces familles et donc c'est une fracture sociale et ce n'est pas juste l'article 36 propose donc de remédier à ces difficultés en déterminant désormais le CMG en fonction des ressources de la famille du nombre d'enfants à charge du nombre d'heures et du coup médian de la garde, dès lors, les taux d'effort des familles Sega liseré à la manière de la participation demandée pour un accueil en crèche relevant de la prestation de service unique du PSU, l'article 36 prévoit aussi la possibilité pour les familles monoparentales, de recevoir le CMG emplois Directs jusqu'au 12 ans de leurs enfants contre six ans pour le droit commun, autre lueur la commission soutient la réforme proposée du CMG qui correspond aux attentes des familles, elle a en outre adopté un amendement visant la suspension sans délai du versement du CMG aux familles, cessant de rémunérer l'assistante maternelle ou la garde à domicile mais il y a un mais l'article 36 suscite plusieurs regrets, à commencer par son entrée en vigueur prévue tardivement pour juillet 2025, d'autre part, il aurait sans doute été possible une évolution du barème, accompagné d'un mécanisme de compensation plus satisfaisant en l'état du texte 43 % des bénéficiaires actuels du CMG seraient défavorisés à l'application de la réforme, qu'est-il proposer à ces familles perdantes l'article prévoit un complément compensatoires aux paramètres incertain et placé sous condition de ressources et au recours minimal aux modes de garde, la réforme se fera donc bel et bien, au détriment de certaines familles déjà déjà engagés auprès d'une assistante maternelle ou d'une garde à domicile, une seconde mesure prévue à l'article 37 oblige l'employeur à verser aux salariés en lieu et place des CPAM une somme au moins égale aux indemnités journalières pour congé de maternité d'adoption ou de paternité, l'employeur serait ainsi su Breger dans les droits des assurés de percevoir les indemnités si certains employeurs ont choisi librement cette option moi applique la la matière, un accord de branche. Une telle obligation légale de versements semble disproportionnée en raison des charges de trésorerie qu'elle fait peser aux entreprises indistinctement de leur taille ou de leur situation, la Commission vous proposera donc de supprimer cette disposition comme vous le constaterez mes chers collègues, de nombreuses autres mesures attendues des familles sont absentes de ce Plfss je pense à la réforme de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, la prépare ou à la fin de la modulation des allocations familiales, selon les revenus, le retour à à l'université, la IT mesure votée par le Sénat en février dernier, il convient aussi de s'atteler à la création de places en crèche. Attendue par les familles, indispensable pour l'égalité hommes-femmes et puis pour ce qui concerne une employée Pellier plus forte, notamment des femmes et aux difficultés de recrutement des professionnels de la petite enfance qui est chaque jour plus important, on parle de 10000 personnes, 10 1000 places disponibles 10000 places attendu toutes ces avancées ne se feront pas sans coût financier, c'est pourquoi nous devons préserver les marges de manoeuvre budgétaires de la CNAF pour une relance véritablement ambitieuse de la politique familiale, je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est maintenant à monsieur Philippe mouiller, rapporteur de la commission des affaires sociales pour l'autonomie, pour cinq minutes. C'est le président, mesdames, messieurs les ministres, madame la présidente de la commission madame le rapporteur général, mes chers collègues annoncé triomphalement par le précédent gouvernement, la nouvelle étape de l'histoire de la sécurité sociale qui était la création de la branche autonomie présente pour le moment un bilan bien mince, le débat sur le périmètre de la branche, hein, et pour l'instant, les assurés n'ont pas vu évoluer les choses, une nouvelle concertation vient de s'ouvrir pour tracer les perspectives du bien vieillir, elle rendra ses conclusions au printemps prochain, au moment où débutera la concertation sur le handicap, il ne faut plus tarder, Monsieur le Ministre, les défis à relever sont connus, les besoins de recrutement ne font que croître et le secteur a besoin de financements supplémentaires environ un degré 5 milliards pour le seul secteur des personnes âgées, l'objectif de dépense de la branche pour 2023 s'élève à 37 vers les 4 milliards d'euros, en augmentation de 5,3 % par rapport à l'année précédente, malgré cet effort, comme l'année dernière, ces hausses résulte principalement des revalorisations salariales mises en oeuvre dans le cas du Ségur de la santé et de son extension à d'autres personnels non médicaux des établissements et services sociaux et médico-sociaux, par ailleurs, je ne peux que regretter que ces efforts budgétaires supplémentaires ne permettent toujours pas de traiter la situation de l'ensemble des oubliées du Ségur agent pourtant indispensables au fonctionnement du secteur, les projections pluriannuelle, indique que la branche autonomie retrouvera une situation excédentaire à compter de 2000 vingt-quatre un excédent qui diminuerait les années suivantes, du fait des 50000 créations de postes annoncées en Ephad et du financement du temps dédié au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficie du plan d'aide à domicile, dans ce contexte, il ne resterait aucune marge budgétaire disponible pour faire évoluer la situation et les conditions de vie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, ce qui est inquiétant aujourd'hui et nous sommes sollicités de partout par les institutions du monde du handicap, qui s'inquiète de cette situation. Lors de votre édition devant la commission, monsieur le Ministre, vous avez parlé d'un PLFSS de fin de cycle, c'est le cas, les dispositifs proposés par le texte Vienne sécuriser des formes, des réformes déjà lancé les années précédentes et renforce le virage domiciliaire qui est la principale orientation stratégique, suivie par la branche attention qui répond à la demande des personnes en situation de perte d'autonomie bien sûr le PLFSS porte la marque des soubresauts qui ont secoué le secteur des Epad à la suite de la publication du livre les fossoyeurs et de la nécessité pour le gouvernement de combler ce que nos collègues Bernard Bonnet et Michel Meunier ont appelé les angles morts du contrôle ces mesures virage domiciliaire contrôles vont dans la bonne direction, elles illustrent ainsi les limites d'une méthode consistant à retoucher ce qui peut l'être en loi de financement, la vision d'ensemble est quasi absente la concertation préalable avec les professionnels ou les départements faible mais la complexité s'accroît à chaque dispositif nouveau songer que les concours de la CNSA au département transiteront désormais par plus d'une dizaine de canaux différents. Ah, ces dispositifs d'intérêt variable, l'Assemblée nationale a ajouté 19 autres articles un record dont on se demande de rapport pour la seule branche autonomie parmi ces dispositions, j'en remettrai trois en exergue la revalorisation annuelle du tarif plancher qui passera à 23 euros en 2023 la création d'un parcours de rééducation de réévaluation des enfants en situation de poulet handicap ou de paralysie sidéral et une expérimentation visant à assurer un meilleur accommodions des aidants toutefois la question du financement de ces mesures nouvelles récentes hier et inquiète les départements qui ne peuvent supporter de nouvelles charges sans aucune visibilité. Aujourd'hui ils ont un dialogue, une discussion, mais pas de certitudes. Un souffle nouveau nécessaire l'engagement de réflexion stratégique sur l'autonomie est indispensable, il faut réfléchir à la création de ressources nouvelles et surtout imposer une vision pluri-annuel qui ne se résume pas à dit non Havre mission et groupes de travail et ce thème pluriannuel est essentielle pour l'ensemble du secteur. Pour maintenir les questions d'autonomie à l'agenda politique quand enfin une vision stratégique soit nourri par des données et que des décisions de financement soient prises, la commission des affaires sociales vous propose d'institutionnaliser le dialogue entre les différents partenaires sous la forme d'une conférence de génération de l'autonomie puisse ces hein sans jouer le rôle qu'à la conférence nationale du handicap pour faire progresser la prise en charge des plus fragiles et très concrètement pour terminer mes propos, je voudrais vraiment, hé bien l'orientation donnée par le nombreux acteurs du secteur qui s'inquiètent, non pas de la prise en compte de leurs préoccupations, mais des délais de la programmation et surtout des moyens nécessaires, avec une perspective d'avenir, je vous remercie de votre attention. Merci, cher collègue là. La parole est maintenant à monsieur Christian Klinger, rapporteur pour avis de la commission des finances pour cinq minutes.

Monsieur le président, Mesdames et messieurs les ministres, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame, le rapporteur général, mes chers collègues, la commission des finances, a constaté que le PLFSS comportait peu de mesures impact financier significatif pour 2023, l'évolution des recettes et des dépenses résulte essentiellement de paramètres inchangé par rapport à cette année, et des hypothèses macroéconomiques retenues par le gouvernement, celle concernant la masse salariale ont été jugé plausible par le Haut Conseil des finances publiques, mais nous savons qu'il existe un aléa sur la prévision de croissance et que des signes de ralentissement apparaissent la prévision de dépenses tablent sur une quasi-extinction des prises en charge dérogatoire liée au Covid 7 moindres dépenses escompté mais incertaine, explique à elle seule, la diminution du déficit de la Sécurité sociale pour 2023 or crise sanitaire, le déficit 2023 sera simplement stabilisé par rapport à 2022 malgré des hypothèses de revalorisation des prestations pour l'an prochain, sensiblement inférieur à l'inflation et à condition de conserver une évolution positive de l'emploi, une bonne dynamique de la masse salariale. Le déficit de l'assurance maladie se réduit fortement, c'est l'effet du faible montant de la provision pour la crise sanitaire s'y ajoute la ponction de 2 milliards sur la branche famille injustifiée et inopportune au moment où le fléchissement de la natalité exigerait une politique familiale plus ambitieuse. Les mesures de maîtrise des dépenses d'assurance-maladie paraissent conjoncturelle plus que structurelle certaines économies attendues sont peu documentée, notamment les actions sur la pertinence des actes et des prescriptions. La commission des finances, relève néanmoins plusieurs dispositions du texte visant à renforcer la lutte contre les abus et les fraudes. Dans l'enquête remise il y a 2 ans à la commission des affaires sociales du Sénat, la Cour des comptes avait dressé un constat sévère sur l'insuffisance des contrôles réalisés par l'assurance maladie, les modifications proposées vont dans le bon sens mais il faudra amplifier ces actions, les prévisions pour 2024 et au-delà nous paraissent inquiétantes à plusieurs titres premièrement, le déficit persiste et s'accentuer à partir de 2000 vingt-quatre alors que les hypothèses de croissance, d'emploi et de recettes sont optimistes, deuxièmement, les prévisions de dépenses d'assurance-maladie, sont elles aussi optimiste avec un rythme d'évolution inférieur à celui de la croissance majoré de l'inflation. Ce résultat supposerait une maîtrise des dépenses particulièrement efficace mais les instruments n'en sont pas véritablement précisé. la trajectoire des dépenses de retraites avec une nette dégradation dès 2000 vingt-quatre et d'autant plus préoccupante que le gouvernement indique avoir en partie prises en compte, à un niveau qui n'a cependant pas clairement précisé les effets d'une nouvelle réforme. Le relèvement de l'âge de départ est désormais jugée absolument hein indispensable alors que l'idée on était totalement écarté en 2017, le Sénat lui a été constant sur ce point en inscrivant depuis 2014 dans chaque PLFSS une mesure dans ce sens. En tout état de cause, cette réforme constamment repoussées sera engagée trop tardivement pour avoir un effet sensible sur le rythme de progression des dépenses de retrait de recettes d'ici 2027, en résumé, le Plfss pour 2023 comporte peu de mesures de nature à rééquilibrer les comptes sociaux, l'amélioration affichés pour l'an prochain n'est due qu'à une quasi-disparition escompté de toute mesure spécifique à la gestion du Covid, les déterminants des déficits persistent et les sont sans doute sous-évalués. Le projet se place en outre dans une perspective de comptes sociaux dégradé durant plusieurs années avec la remontée des déficits dès 2024, la question de leur financement se posera donc inévitablement d'ici 2 ans quand les possibilités de reprise par la qu'auront été épuisés dans un contexte de taux sans doute plus difficile que celui de ces dernières années. Pour ces raisons, la commission des finances, a considéré que le projet de loi n'était pas acceptable en l'état, elle a donc conditionné son avis favorable à l'adoption des amendements présentés par la commission des affaires sociales, dont elle partage pleinement l'objectif je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est maintenant à Madame Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales pour cinq minutes. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les Ministres, madame la rapporteure générale, mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 et le premier que nous examinons sous l'empire d'un cadre organique rénové, celui-ci était censé en particulier améliorer nos délais d'examen et renforcer l'information du Parlement, je crois que nous n'avons jamais connu délais d'examen aussi court et dégradé et je voudrais rendre hommage à nos rapporteurs qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour présenter à la Commission, puis au Sénat, une position cohérente sur ce texte, quant à l'information du Parlement, nous aurons sans doute encore à y travailler, la loi organique ne suffisant pas à parvenir aux objectifs fixés sur le fond, nous aurions pu attendre dans les circonstances de l'engagement de la responsabilité du gouvernement un texte resserré sur l'essentiel, traçant quelques axes stratégiques pour l'avenir de la sécurité sociale le 49 3 ne nous aura pourtant pas épargné un texte bavard, dont le volume a encore une fois plus que doublé, été non seulement de quelques fonds de tiroir de ministères, mais aussi de demandes de rapport, nombreuses dans les faits concrets sur le cours des choses et inversement proportionnelle à l'émotion suscitée par leur adoption je n'évoquerai pas dans le détail des dispositions certes sympathique, mais dont la place dans le texte n'est pas toujours évidente, c'est sans doute qu'il demeure un malentendu assez fort sur ce qui nous occupe aujourd'hui le PLFSS n'est pas le lieu d'une discussion prospectif sur notre système de santé ni même sur l'organisation de notre protection sociale en général, il devrait être un des points d'orgue de notre vie démocratique, le moment où gouvernement et Parlement justifie devant nos concitoyens du bon emploi des sommes qui leur sont demandés pour le financement de la protection sociale, rappelons que nous allons franchir l'année prochaine le cap symbolique des 600 milliards d'euros de dépenses, c'est bien plus que le budget de l'État, c'est bien plus que le financement d'autres politiques publiques qui ont toute leur importance, que l'on songe à la Défense à l'éducation, la recherche ou encore à la justice pour n'en citer que quelques-unes dans un contexte où les Français souffrent de la hausse des prix et de conditions de vie de plus en plus difficile, nous sommes ici pour justifier des prélèvements sur le revenu pour leur assurer une protection solidaire, en effet, malgré les sommes très importantes qui lui sont consacrés, notre modèle social est en crise structurelle l'hôpital semble en plus mauvaise posture qu'au plus fort de la crise, l'accès aux soins souffrent d'inégalités insupportables, qu'elles soient sociales ou territoriales, les retraites sont mises à l'épreuve de la démographie et nous abordons, non sans inquiétude, mais dans l'impréparation, le mur de la dépendance de génération du papy-boom devant une protection sociale dont le modèle solidaire et menacé que nous propose ce texte un statu quo un peu incompréhensible puisque le tableau d'équilibre avant mesure nouvelle est identique à celui d'après mesures à ceci près que les dépenses nouvelles sont venues aborder les recettes nouvelles nous sommes responsables devant les Français de l'efficacité de la dépense publique et de la préparation du pays aux défis de demain, c'est à cela que nous devrions consacrer nos débats d'aujourd'hui comment sortir d'une économie de crise : comment faire face à l'inflation à la remontée des taux d'intérêt alors que la dette sociale ça accumulé comment accueillir l'innovation et favoriser le vieillissement en bonne santé, nous n'avons trouvé aucune réponse à ces questions dans le PLFSS néanmoins en responsabilité, porté par l'exigence que nous devons aux français par un attachement profond à la soutenabilité de notre modèle social pour pouvoir le laisser aux générations futures, la commission des affaires sociales, vous en proposera quelques-unes, elle passe par une adaptation de notre modèle aux défis du moment mais aussi un renforcement de la reddition des comptes du gouvernement devant le Parlement, et à travers lui à l'ensemble de nos concitoyens, je vous remercie. Nous passons maintenant à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable mesdames, Laurence Cohen, Katia pour se et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste ont déposé une motion distribuée sous le numéro 762 tendant à Pau à opposer la question préalable en textes en discussion, la parole est à madame Laurence Cohen pour la motion pour dix minutes. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les ministres, madame, le rapporteur général, mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues permettez-moi de citer le gouvernement lors de la présentation, le 23 septembre dernier de ce budget de la Sécurité sociale pour 2023 en sortie de crise sanitaire et en début de quinquennat ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale est un texte d'ambition pour répondre aux enjeux du quotidien des Français pouvions-nous croire que la crise sanitaire et la crise du pouvoir d'achat de nos concitoyennes et concitoyens vous ferait changer de logiciel libéral, le gouvernement les-t-il enfin arrêter d'épuiser les recettes de la Sécurité sociale avec les exonérations de cotisations patronales, que nenni le PLFSS 2023 prévoit une augmentation de 5 milliards d'euros des exonérations sociales patronales pour atteindre 70 milliards d'euros en 2023 le gouvernement allait-il enfin prendre en charge ses responsabilités en assumant la dette de la cadette de 18 milliards d'euros de la pandémie de Covid un amendement du groupe communiste à l'Assemblée nationale avait d'ailleurs été adoptées pour transférer la dette du budget de la Sécurité sociale vers le budget de l'État au contraire le gouvernement actionné à 2 reprises l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour passer outre l'opposition parlementaire et au passage à supprimer cette disposition pour débattre, mes chers collègues, il faut en avoir la volonté politique, or elle n'est pas au rendez-vous, loin s'en faut, monsieur le Ministre, vous refusez d'antan de la souffrance des personnels des secteurs de santé et du médico-social, celle des patients qui n'ont plus de médecin traitant ou qui attendent des heures sur les brancards dans les couloirs des hôpitaux en persévérant dans vos choix en amplifiant la logique qui est la vôtre, qui considèrent la santé comme un coup qu'il faut réduire, vous détruisez la sécurité sociale à laquelle les Françaises et les Français sont tellement attachés et vous précipiter les départs des hospitaliers, la situation est critique et annonce un point de non-retour, pourtant vous persévérez signé une politique irresponsable en prévoyant une progression des dépenses de l'assurance maladie à seulement 3 7 % mais en réalité, en diminution de 0,8 % en tenant compte de la crise sanitaire, le budget de la santé va augmenter moins vite que l'évolution naturelle des dépenses de santé, de 4 l'Ondam va demeurer un point en dessous de l'inflation estimée à 4 7 % pour 2023, ce qui est une première bien funeste, hein, si vous allez réaliser 1 virgule 7 milliards d'euros d'économies en 2023 sur le budget de la santé, autant d'argent qui va manquer pour recruter du personnel donc améliorer leurs conditions de travail, interrompant l'hémorragie du personnel qui n'en peut plus pire vous justifier les fermetures de lits 21000 lits, entre 2017 et 2 1000 22 et de service par manque de personnel, mais à qui la faute, qui refuse de donner des moyens supplémentaires aux universités qui ne réintègre pas les personnels licenciés durant le Covid, qui ne prend pas en charge les formations, laissant les hôpitaux se débrouiller vous attendez la montée des colères pour débloquer quelques millions cent vous en prendre à la racine des maux de notre système de santé, le manque de recettes volontairement entretenu quand une maison menace de s'effondrer, pensez-vous que l'urgence est de repeindre la façade, c'est pourtant ce que vous faites au gouvernement, je pense notamment à la situation des services pédiatriques sur laquelle je vous ai interpellé lors des questions d'actualité, Monsieur le Ministre, le 26 octobre dernier, là encore, vous m'avez opposé une fin de non-recevoir, balayant l'effet que je reporter d'un revers de main, pourtant je ne faisais que relayer la colère, l'indignation des principaux intéressés, écoutez le préfet, le professeur Stéphane Dauger, chef de service de réanimation pédiatrique de l'hôpital Robert Debré qui ne décolère pas, lui non plus, entendent que tout est sous contrôle ça relève presque de la provocation pour ceux qui, sur le terrain se confronte à cette crise, dit-il, même en travaillant jusqu'à l'épuisement, on doit refuser des patients, alors que les personnels de la pédiatrie dénoncent depuis des années les manques de moyens humains et financiers, le gouvernement a jugé suffisant d'accorder une prime de soins critiques et le doublement des heures de nuit mais uniquement jusqu'au 31 mars 2023, l'épidémie de bronchiolite n'est que le sommet de l'iceberg de la réalité des urgences pédiatriques qui cours tout le reste de l'année, le déblocage de 400 millions d'euros, est une insulte pour les personnels mobilisés, d'autant que 150 millions étaient déjà prévues pour l'ensemble des services en tension de l'hôpital, les services pédiatriques, comme l'ensemble des services des hôpitaux ont besoin de mesures structurelles pour pallier aux conséquences des politiques d'austérité menées par les différents gouvernements qui se sont succédé depuis près de 20 ans, les difficultés d'accès aux soins rencontrées par nos concitoyennes et nos concitoyens nécessite de recruter 100000 personnels dans les hôpitaux et d'augmenter les capacités de formation des universités pour former d'davantage de médecins mais aussi de paramédicaux comme les infirmières et les infirmiers qui subissent des conditions dégradées de formation dans les IFSI au lieu de ces mesures d'urgence, urgence, vous préférez ajouter une dixième année aux internes de médecine et privé les territoires d'une génération de médecins en 2026 cette réforme s'est faite sans consultation des organisations syndicales des internes ni réflexion sur le contenu pédagogique, alors que tout récemment, les études de médecine, on subit de profondes réformes dont les effets n'ont pas encore été évalués, vous allez réduire l'attractivité de la formation de médecine générale, le gouvernement, tout comme la majorité sénatoriale ne sont pas en phase avec l'aspiration des jeunes générations qui souhaitent exercer dans des structures collectives en étant salarié pourquoi refusez, Monsieur le Ministre, de financer les centres de santé à la même hauteur que les maisons de santé où les médecins libéraux, pourquoi un centre de santé doit se contenter d'une aide financière à l'installation de 30000 euros quand les maisons de santé, les médecins libéraux bénéficient eux de 50000 euros la création de Centres de santé, pourtant l'une des réponses pour combattre les déserts médicaux et paramédicaux qui s'étendent sur tout le pays, pourquoi ne pas avoir le courage de rétablir les gardes de médecin, le soir, le week-end et les jours fériés pour ce faire, il y aurait urgence à revaloriser le montant des gardes et à étendre cette obligation à l'ensemble des médecins généralistes, y compris en secteur de au lieu de ces mesures de bon sens de justice qui nous remonte des établissements hospitaliers de nos territoires, des syndicats, des collectifs, vous choisissez d'exonérer de cotisations sociales, les médecins retraités pour qu'ils poursuivent leur activité, on marche sur la tête ce PLFSS c'était l'occasion de tirer des enseignements de la pandémie et des incertitudes, des conséquences de l'apparition d'un nouveau variant, comment ne pas être en colère de constater Monsieur le Ministre, que pour le financement des tests et des vaccins Covid vous n'avez provisionné seulement qu'un milliard pour 2023 quand les mesures d'urgence sanitaire ont ont coûté plus de 11 milliards en 2022 à l'assurance maladie, alors que l'espérance de vie en bonne santé de 64 ans dans notre pays, le gouvernement et la majorité sénatoriale souhaite reculer, reculer l'âge légal de départ en retraite à 64 ans, plutôt que d'augmenter les cotisations patronales de quatre euros par mois pour assurer le financement des retraites de cette réforme, nous n'en voulons pas ce PLFSS c'était l'occasion, à défaut d'une grande loi grand âge annoncé à maintes reprises de s'engager sur la voie du recrutement de 100000 paires professionnels par an pendant 3 ans pour les Epad afin de parvenir à un encadrement d'un résident par un soignant, on est loin 70 millions d'euros pour recruter dans les EPHAD représente un demi-poste de plus dans chacun des 7000 et pas de France après le scandale Orpea allez-vous continuer à laisser des organismes à but à but lucratif, gérée massivement les établissements qui accompagne nos ennemis allez-vous continuer à les laisser faire des profits sur leur dos, on le voit, Monsieur le Ministre votre projet pour accompagner nos anciens est un projet de société, aux antipodes de celui que je porte avec un groupe, je parlais au début de mon propos d'étatisation de la Sécurité sociale et de sa remise en cause, ce constat se confirme par le transfert à la branche famille des indemnités journalières des congés de maternité post-naissance jusqu'ici pris en charge par l'assurance maladie, en fait, en conclusion, je peux dire monsieur le ministre, et messieurs, mesdames les ministres, ce que ce budget est totalement déconnecté de l'urgence, il est injuste, pour ne pas dire provocateur inégalitaire et sincère, alors que le Sénat doit examiner en quatre jours un budget de 600 milliards d'euros, je rappelle que le projet de loi de finances et d'examiner sur trois semaines pour un budget de seulement 480 milliards d'euros, alors que le gouvernement a utilisé le 49 3 à 2 reprises à l'Assemblée nationale, le Sénat a utilisé son 49 3 interne en déclarant irrecevable la moitié des amendements déposés sur ce PLFSS dimanche le président du Sénat, déclarait pourtant dans le journal Le Parisien que le Sénat disputerait sur le fond de tous les sujets, le soir même, la commission des finances, a jugé irrecevable des amendements, comme la mise à contribution des entreprises responsables d'accidents médicaux au financement de la branche accidents du travail et je cite l'argument parce qu'il vaut son pesant de cacahuètes si je puis m'exprimer ainsi, l'amendement a un effet trop indirect et incertain sur les finances de la Sécurité sociale, cette censure du Sénat et le coup de force démocratique du gouvernement démontre l'absence de volonté de débattre réellement des propositions alternatives de l'opposition pour l'ensemble de ces raisons, les sénatrices et les sénateurs du groupe communiste républicain citoyen écologiste invite tous les parlementaires attachés à la sécurité sociale solidaire universel et financée par les cotisations à voté notre motion, je vous remercie. Merci, cher collègue. à l'heure, quel est l'avis de la commission sur cette motion. Merci, cher collègue, pour l'ensemble de, de, de votre prise de parole parce que, en réalité, ça me donne l'opportunité de de vous dire que finalement il y a beaucoup d'appétence chez vous à vouloir débattre et là ce que vous proposez c'est de couper court au débat sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, c'est l'argument facile plus loin pour aller plus loin, madame la présidente, la réalité c'est que, effectivement, vous êtes le porte-voix d'insatisfaction et que sans doute il faut aussi les porter au gouvernement mais c'est une opportunité de débattre de chaque article de chaque amendement et de pouvoir justement porter ces difficultés que dont vous avez connaissance sur le terrain et donc moi je vous encourage beaucoup plus, a, finalement, ne pas voter cette motion pour justement que nous puissions avoir ce débat d'autant plus que ce débat n'a pas eu lieu à l'Assemblée nationale dans sa totalité, en tout cas, donc c'est un avis défavorable de la commission. Merci, merci, merci, la parole est au gouvernement pour son avis, monsieur le Ministre. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, avis défavorable pour me donner la possibilité, justement, de débattre sur les sujets de santé. Merci, monsieur le Ministre, y a-t-il des explications de vote Monsieur Jomier Madame mange. Merci monsieur le président, au nom de mes collègues, que si nous votions avec notre coeur nous voterions probablement la question préalable de nos collègues communistes parce que beaucoup des arguments et pas seulement le 1er avancé par Laurence Cohen sont justes. Et en particulier les conditions d'examen de ce texte. C'est rare qu'un PLFSS arrive au Sénat à la suite d'un 49 3 à l'Assemblée nationale, certains pour nous dire quand c'était la dernière fois, je ne le sais pas mais en tout état de cause, c'est la première fois, dit la rapporteure générale, en tout état de cause, arrive un test qui n'a pas été débattue complètement et qui mérite donc qu'on le débat à fond et sereinement et je dois dire qu'à cet égard le 49 3 ben rend incertain nos délibérations par essence puisqu'on sait que quand elle repartira à l'Assemblée nationale, il sera l'objet d'un nouveau 49 3 donc on ne sait pas trop s'il est très utile de mener certains débats et deuxièmement parce que dans la gestion des irrecevabilité la majorité sénatoriale n'a pas simplifier notre tâche et que, encore une fois, je m'inscrirai dans les pas de très respecté Jean-Pierre Sueur pour dire et je l'ai constaté que des amendements qui était recevable l'an dernier, ne le sont plus cette année et que la lecture par les différentes commissions du régime des hérésie recevabilité nous empêche de mener au fond, certains débats nous contraint à utiliser des artifices que qui sont des artifices, les demandes de rapport et cetera et que tout Sami Abou fait que ce budget de la Sécurité sociale va être débattue dans des conditions dégradées pour autant nous nous abstiendrons pour débattre mais il n'y avait pas qu'un seul argument du groupe communiste, qui était recevable, je vous remercie. Oui, merci Monsieur le Président, alors effectivement nous nous partageons avec le groupe CRCE le constat sur le PLFSS qui est loin de répondre aux défis qui sont les nôtres, un Ondam, encore une fois, insuffisant, notamment hospitaliers qui oblige encore à des économies, alors que la situation de l'hôpital public est plus que critique des pans entiers du soin sont tout simplement oublié, rien sur la psychiatrie, rien sur l'apéritif il est insuffisant sur l'autonomie il est insuffisance sur la famille, et en plus, les mesures sont reportées en fait je tout de suite venir aussi ou c'est un PLFSS sans souffle, hein, qui perpétue une lente désagrafé désintégration du système de santé par une gestion comptable de court terme arriver effectivement par le 49 3, nous ne sommes pas assuré d'ailleurs que ce PLFSS ne ressorte de nouveau à l'Assemblée nationale, plus tard, de la même manière antidémocratique et là je confirme effectivement qu'il y a dans les les motifs d'irrecevabilité des choses c'est l'Arctique quarante ça hein du ça a un impact sur les recettes de la Sécurité sociale, mais il y a beaucoup d'amendements qui ne sont pas pris parce qu'ils n'ont pas d'impact sur les ressources ou les dépenses de la Sécurité sociale, alors je, je dirais que quelque part c'est un peu paradoxal, nous reproche d'avoir un impact notamment négatif, bien sûr, soit effectivement d'avoir un impact insuffisant ou indirect ou mal contrôlés moi l'évoluer sur sur la protection sociale, il y a effectivement un abus aujourd'hui des irrecevabilité merci. Merci, je vais consulter le Sénat sur la motion Merci monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente, madame, le rapporteur général, mes chers collègues, donc si vous voulez, on peut pas dire que l'Ondam, n'a pas augmenté puisqu'il a augmenté de 57 milliards depuis 2017 alors actuellement il y a un manque de médecins, c'est vrai qu'on peut trépigner des pieds, mais malheureusement il y en a pas, il y a eu le effectivement le numerus clausus, qui a été modifiée, mais bien sûr ça va on va attendre dix ans, donc il y a eu aussi le Covid quand même, il faut dire que ça quand même perturber beaucoup, la sécurité sociale, il faut quand même rappeler les 35 milliards de déficit en 2020, alors je pense que dans ce PLFSS il y a des choses qui sont très valables de progrès comme les inciter effectivement les médecins retraités à pouvoir continuer leur activité, inciter les médecins à participer au service d'accès au sein et à la régulation

être dans le médico-social et ça c'est très important, vous nous avez dit que ça allait arriver, mais c'est vrai que nous ne vont pas oublier ce pro cette ces progrès qui a dans P2P, certes le dépistage sexuellement sexuellement transmissibles, c'est très important pour la stérilité des grossesses extra-utérines les vaccinations avec les pharmaciens, les infirmiers, les sages-femmes, c'est très, c'est aussi très important, les consultations aux âges de la vie aussi la contraception d'urgence pour toutes les femmes, c'est quelque chose de très important et les efforts pour les familles monoparentales, donc pour les français, je pense que nous devons examiner ce PLFSS améliorer merci.

lors de la discussion sur les amendements de d'en discuter, d'en débattre, mais plutôt sur la motion préalable et dire que notre groupe est attaché au débat la démocratie c'est la discussion c'est le débat la motion préalable si on l'a voté, ce sera en quelque sorte un 49 3 à l'envers parce que, imaginez que l'Assemblée nationale adopte les textes, ce texte en 49 3 que nous on voterait cette motion préalable et je pense que ce serait tout simplement la la négation du Parlement et et même en quelque sorte du Sénat, donc, pour une raison d'attachement à la démocratie et parce que aussi, nous sommes impatients, même quand nous ne sommes pas d'accord, nous sommes impatients, même quand nous ne sommes pas d'accord, d'écouter vos vos arguments, je pense que nous avons la responsabilité de de débattre de ce PLFSS je vous remercie. Oui, Monsieur le Président, compte-tenu des enjeux, je pense qu'on ne peut que débattre en plus un amendement peut être, je veux dire le 49 3 ne n'empêche pas pour autant que la loi puisse progresser, évoluer, donc je crois qu'il est extrêmement important eu égard, encore une fois à l'importance des enjeux et au sujet qu'on va traiter ne serait-ce que par respect pour les Français, de montrer que le Sénat, travaille, travaille de manière constructive. Merci, pas de regret c'est parfait. Je vais consulter le Sénat sur la motion tendant à opposer la question préalable, je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du texte en discussion en application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire et de droit, le scrutin public est ouvert.

plus personne ne demande à voter. Cette fois-ci, plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos.

Sur la motion 762 compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordé par les sénateurs groupes politiques et notifié à la présidence Nombre de votants : 344 Nombre de suffrages exprimés 278 pour l'adoption 27 contre 251 le Sénat n'a pas adopté. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à madame Chantal de scène pour le groupe Les Républicains pour huit minutes, vous, vous avez la parole, ma chère collègue. Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente, madame la rapporteure générale ce premier Plfss du quinquennat montrent une amélioration des comptes en trompe l'oeil et temporaire, basé sur des hypothèses économiques optimistes PIB à 1 pour 100 masse salariale à 5 pour 100 et des dépenses de santé sous-estimer le déficit initial de la sécurité sociale fixé à l'origine à 6,8 milliards est passé à 7,3 milliards ne manque une stratégie ambitieuse de réduction des déficits, d'après les prévisions de recettes inscrites à l'article 3 le solde de la branche famille devaient être excédentaire à hauteur de 2,6 milliards d'euros au titre de l'année 2022 mais au travers d'un tour de passe-passe budgétaire : nous assistons à un transfert de plus de 2 milliards au détriment de la branche famille pour améliorer le solde de la branche maladie fortement déficitaire, les dépenses d'assurance-maladie sont donc artificiellement allégées, je rappelle que la bonne situation financière de la branche famille s'est faite au prix d'importantes mesures d'économie qui ont impacté directement le budget des familles dans la continuité du quinquennat de François Hollande, votre majorité rabote chaque année, la politique familiale, notre système de politique familiale, a perdu sa vocation universaliste cette orientation est une grave erreur au moment où les familles subissent de plein fouet une baisse drastique de leur pouvoir d'achat, je déplore également un manque de réformes structurelles, l'absence d'une loi sur le grand âge et le manque de nouveaux moyens financiers montrent que les crédits supplémentaires accordés à la branche autonomie ne sont qu'une rustine sur un système à bout de souffle, chaque année on nous promet une loi sur le grand âge et l'autonomie pour la renvoyer ensuite aux calendes grecques, or, d'après les projections effectuées par l'Insee, là par des seniors de 65 ans et plus, va augmenter de 33 % entre 2000 22 et 2041 puis de 51 % d'ici 2000 70, il est urgent d'anticiper cette évolution démographique, enfin, nous estimons que l'Ondam ne sera pas tenable, comme la développer Corinne Imbert précédemment l'Ondam est en hausse de 3,7 pour 100, mais c'est sans tenir compte de l'influence de à 4 7 % ni de la hausse tendancielle des besoins de santé estimée à 4 % par la commission des comptes de la Sécurité sociale, certaines mesures que vous proposez vont dans le bon sens, tels que la réforme du complément mode de garde allocation perçue par les parents faisant garder leur enfant par une assistante maternelle, une micro-crèche une garde à domicile ou encore une garde partagée. Dans ses intentions, cette réforme est une mesure de justice et d'équité, toutefois, dans sa forme actuelle, elle risque d'abaisser les aides versées à 43 % des familles concernées, c'est inacceptable, qui plus est, au moment où les familles subissent la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation, cette réforme du CMG doit éviter de faire des familles perdantes lorsque la garde d'enfant est indisponible trop cher de nombreuses mères risquent de décrocher de l'emploi mieux soutenir les familles, c'est soutenir l'égalité hommes-femme. Attention aussi à ne parents de la gare trop coûteuse pour les familles faisant gare garder leur enfant à temps partiel, que ce soit du fait du travail à temps partiel d'un parent ou de l'utilisation d'une gare de de santé ce nos politiques de santé se résume souvent à une approche curative la prévention doit être renforcée ce PLFSS propose la mise en place des rendez vous de prévention de l'objectif est de renverser renforcer l'intervention des professionnels de santé, mais concrètement, comment allez-vous organiser ces 3 rendez-vous aux différents âges de la vie, alors que l'on a déjà du mal à trouver des professionnels de santé, en outre, ce n'est pas forcément l'âge de la personne qui doit définir la période de dépistage mais plutôt ses antécédents médicaux. En matière de prévention je je souhaite également attirer votre attention sur la première épidémie non infectieuse de l'histoire de l'humanité, je veux parler de l'obésité en 2012, le ministère de l'Économie estimait déjà à 20 milliards d'euros le coût social du surpoids comparable à celui du tabac ou de l'alcool. Il est regrettable que ce PLFSS ne porte aucune mesure de prévention contre l'obésité dont le coût est si important, enfin, Monsieur le Ministre, je souhaite appeler votre attention sur un tout autre sujet, il s'agit de l'illectronisme en santé, l'illettrisme numérique résulte de l'inaptitude d'un individu à utiliser les outils numériques du quotidien ce phénomène touche 17 % de la population soit presse près de 13 millions de personnes de personnes en France, selon une enquête du monde, 67 2 pour 100 des patients de 75 ans et plus, sont concernés et 43 % d'entre eux sont non diplômés, ces patients victimes de la fracture numérique sont souvent issus de milieux défavorisés et vivent dans des territoires périphériques éloigné du service public hospitalier ne pas pouvoir accéder aux solutions de télésurveillance médicale et pour eux une sorte de double peine, la télé-surveillance a démontré sa pertinence durant la crise sanitaire permettant la continuité des soins sur des pathologies chroniques, elle est aujourd'hui indispensable dans notre territoire et touché par les déserts médicaux et frappé par une pénurie de spécialistes, le dispositif actuelle se concentre sur le remboursement des seules solutions technologiques et écarte par conséquent le suivi humain seul adapté aux patients en situation d'électronique nous devons penser à des solutions pour développer l'accompagnement au digital dans le secteur de la santé, cela fonctionne déjà dans le secteur des associations qui accompagnent les personnes électronique, ce n'est pas très compliqué à mettre en oeuvre, mais la difficulté porte sur les moyens nécessaires afin de lutter plus efficacement contre un système de télé-suivi à 2 vitesses, une partie du budget alloué à la télé surveillance pourrait être fait fléché vers des solutions qui rendre le télé-suivi accessible à tous, ce PLFSS manque d'ambition d'une vision pour l'avenir de notre système de santé le premier PLFSS du quinquennat il est un renoncement à Rochefort, à réformer en profondeur notre système de santé et laisse encore de côté une partie des Français, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à Monsieur Daniel Chassain pour les indépendants pour six minutes. Monsieur le président, Mesdames, messieurs les ministres, madame la présidente, mais madame la rapporteure générale, mesdames et messieurs, rapporteur d'un président de commission, mesdames, messieurs, mes chers collègues, donc je voudrais d'abord dire que dans ce PLFSS l'Ondam augmente de 3,7 % de 141 milliards plus 57 milliards depuis 2017 bien sûr, on a l'inflation qui va rogner un petit peu ça avec l'énergie et et les achats, mais il faut reconnaître que depuis une puis 2020, il y a une augmentation des salaires très important de ce Plfss, prévoit un déficit ramené à 6,3 milliards d'euros comme 18 milliards en 2022, mais seulement 1 milliard pour le Covid, je voudrais d'abord saluer le travail des soignants à l'hôpital et le médico-social, la prévention coup apporte des progrès dépistage IST vaccination contraception d'urgence 3 consultations aux âges clés de la vie est fort pour les familles monoparentales concernant l'accès aux soins,

il les oublier et puis pour l'investissement, l'hôpital est en difficulté depuis longtemps ces médecins et infirmières qui manquent pour prendre des postes non pourvus numerus clausus, c'est des résultats dans 10 ans il faut massivement des aides soignantes, infirmières pour le médico-social et l'hôpital, encourager les médecins participent la régulation, c'est bien aux urgences accueillent des patients peu grave dans une salle à un moment et ouvrir des lits, quand c'est possible, bien sûr,

mais seulement de 3000 postes de soignants en EPHAD c'est insuffisant au vu l'augmentation de la dépendance, le géant moyen pondéré est à 730 nous avons zéro 3 équivalent patients par pensionnaire, il en faudrait 05 ça fait 35000 emplois. soit des Français, on souhaite rester à domicile jusqu'à la fin, hein, vous proposez de créer des heures supplémentaires d'appart et 34 pour plus moins social, c'est bien, mais il faudra un budget dépendance pour aider les départements, vous proposez l'augmentation des places de Ssiad pendant le quinquennat c'est indispensable 240 millions d'euros, cette un bon début pour le virage domiciliaire, tout cela doit se concrétiser par la mise en place du grand âge différée par le Covid hé bien sûr, on peut le comprendre et je sais très bien, Madame la Ministre, que le financement ben ça vient par l'emploi et les cotisations, Monsieur le Ministre, vous devez fixé un objectif pour financer des 50000 emplois le plus vite possible pour la prise en charge de la dépendance, dans le secteur du handicap vous proposer la création de places, détection des TSA, mais je crois qu'aussi faut renforcer pour l'inclusion notamment le maintien des ASH pendant le repas et l'interclasses en ce qui concerne les zones sous-denses il y a 6 millions de personnes qui n'ont pas de médecin traitant, l'article 23 instaure une 4ème année d'internat de médecine en autonomie supervisée qui a poussé des internes, descendre dans la rue, nous devons Monsieur le Ministre, les écouter, quant à la rémunération je sais classe doit se faire par décret, mais pour moi, un médecin junior en dixième année peut remplacer et doit percevoir au minimum dix consultations par jour ça fait 50000 55 1000 euros pour 20 jours de travail, nous pensons que les médecins retraités qui poursuivent leur activité à leur cabinet doivent pouvoir s'ils le souhaitent être maître de stage, j'ai fait un amendement dans ce sens mobiliser les médecins retraités en exonération des cotisations de la came, c'est une mesure juste l'article 24, apporte des aides conséquentes à l'installation, malheureusement, ça ne suffit pas, j'ai déposé un amendement qui paraît utile pour un médecin qui s'installeraient en zone hyper dense peu contraignant, la téléconsultation n'est pas un miracle, notre excellente rapporteure Corinne Imbert le disait, mais malgré tout je pense que dans les zones sans médecin avec une cabine, souvent installés d'ailleurs dans ce local de la pharmacie, c'est un plus, les pharmacies ont joué un rôle très important pendant le Covid et vous en vous êtes vous étendez comme pour les infirmières, les compétences pour la vaccination pour moi, c'est très bien, non, monsieur le ministre, dire un mot sur les pharmacies si vous avez une cystite s'enfièvre le samedi après-midi ou une gastro entérite du nourrisson, le pharmacien ne sera pas rémunérée pour l'instant s'ils délivrent de la fausse homicide de la diarrhée ou du Tiorfan sera pas remboursé par l'assurance maladie, alors que c'est le seul professionnel ouverte, sauf les urgences, il est de même pour le sevrage du tabac, il faut encore améliorer la convention avec les pharmacies ce PLFSS apporte des avancées prévention vaccination mode de garde, mesdames et messieurs les ministres, malgré les difficultés de la sécurité sociale due au Covid, vous devez avec votre expérience, fixer un cap pour l'hôpital urgences psychiatriques pédiatriques pour le médico-social, le plan grand âge pour pour la rémunération des médecins Junior pour mobiliser des médecins retraités pour former massivement aides-soignantes, infirmières, pour plus d'terme au CHU pour apporter plus de pragmatisme au pharmacien. Avec les pharmaciens concernant les retraites, à titre personnel, je voterai l'amendement de Monsieur René Paul Savary pour équilibrer conserver les retraites par répartition qui sont en déficit pour le régime de base de près de 16 millions en 2026 cet amendement appel à renforcer l'action des partenaires sociaux avec des propositions de l'accélération de la loi Touraine report à 64 ans, ça c'est des partenaires sociaux qui qu'on en tenant compte des métiers pénibles et mobilisation pour l'emploi des seniors, monsieur le Président, je finis merci. je finis merci. C'est toujours un bonheur déjà l'année dernière j'ai présidé la discussion générale sur le PLFSS moi qui suis un inquiet permanent, hé bien, c'est bien comme débat à toutes les maladies sont possible, même le week-end. Allez. La parole est à Madame Raymonde Poncet mange pour le groupe écologiste pour six minutes. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues. Des années durant, la France fut envié pour son système de santé aujourd'hui, on observe des risques d'effondrement notamment. Son hôpital public des urgences sont déserts médicaux : le système de santé repose désormais sur les dernières forces du personnel en sous-effectif chronique et qui après la politique active de fermeture du gouvernement des gouvernements successifs assistent impuissants aux fermetures de lits place et berceau par manque de personnel, 1000 berceau pour les crèches du Rhône jusqu'à 20 % des places du centre de cancer Gustave-Roussy et la psychiatrie et la pédiatrie sinistrés penser la moitié des lits à Necker de neurochirurgie pédiatrique sont fermés six ans durant les PLFSS annuel se sont sans programmation pluriannuelle de financement que supposerait une vision à long terme de la loi autonomie à une grande loi de santé réclamée par tous les acteurs de santé hospitalier de ville passer l'été passé l'hiver et demain de nouveau l'été ne fait pas une politique, et seul un horizon d'amélioration radicale de notre protection sociale en lui allouant des moyens en conséquence peut enfin redonner sens à l'effort, du personnel et mettre fin à sa désertion au lieu de cela les Budgets sucer successifs valide un Ondam de pure maîtrise comptable qui maintient le système en asphyxie financière suite à une politique organisé organisé de mise en déficit des causes des comptes sociaux à coups d'exonérations de cotisations, loin d'être toute compenser d'exception d'extension, d'assiettes, touchant près aujourd'hui de 10 pour 100 de la masse salariale privée et ce, alors que les besoins sont en progression, le gouvernement et ce qui c'était cette critique en présentant un Ondam hospitalier à 4,1 pas pris, on a pris en compte que 2 tiers de l'indice hospitalier de l'inflation estimée à 5,4 % soit manquant un point dont dame est pas tous les surcoûts Covid et, d'après le calcul unanime des fédérations hospitalières, il manque un milliard avec l'inflation notamment, et une évolution mécanique à 4 % du à la transition démographique à la progression des maladies chroniques, le compte n'y est toujours pas et l'écart des limites et l'écart des limites les économies exigées, même en l'absence de la dite ligne d'économie avec ce sous-financement chronique de l'Ondam se poursuit la destruction de l'hôpital public assis sans revalorisation de l'indemnité de suggestions et du temps de travail additionnel pérenne les professionnels continueront à déserter l'hôpital l'intérim prospérera et la loi risque accélérera de fait, la fermeture des services publics et privés non lucratifs sur chaque, l'heure est un choc d'attractivité par des employes valoriser permettant un travail de qualité auprès de tous les publics, comment peut-on se tromper de diagnostic, on ne voyant pas le problème du côté de la qualité des emplois, alors que 20 % des places ne sont plus remplies en deuxième année de formation sage-femme que 10 % des. étudiant en médecine abandonnent en cours des d'études que des secteurs entiers font face à des démissions, alors qu'il n'arrive plus à recruter la détérioration continue des conditions de travail engendre un sous-effectif qui dégradent à nouveau les conditions de travail et les secteurs entrent dans un cercle vicieux qui pourront sortir suppose de l'ambition, ce que, par exemple, l'objectif de 3000 créations de postes en est pas ne porte pas quand il en faudrait 6 fois plus chaque année, face à la transition démographique au virage, hier, nous prenons un grave retard dans la prévention de la perte d'autonomie, et comme pour la transition écologique ce retard nous coûtera plus financièrement bien sûr, mais ici en espérance de vie en bonne santé, aujourd'hui 20 % des plans d'aide à pas et PCH ne sont pas effectif, faute de personnel, un dossier sur 5, voire un sur quatre restent en souffrance et selon la Cour des comptes, des millions de journées de travail sont perdues tous les ans, du fait d'accidents du travail dans les c'est pas du off au faible ratio d'encadrement cette sinistralité exceptionnelle en est pas s'inscrit dans un contexte où la France, c'est la plus mauvaise élève en Europe en matière de morts liés activité professionnelle or tandis que 1200 personnes meurent tous les ans la branche AT-MP ton excédent et même après transfert à la branche maladie du fait de la soupe et ceci même après ce transfert du fait de la sous-avez sous-évaluation des AT-MP qui prive, rappelons-le, les salariés des droits afférents, la Confédération syndicale européenne exhorte les États à s'engager pour 0 mort au travail en 2030, voilà de quoi utiliser au mieux les excédents nous saluons les mesures en faveur des familles monoparentales, nonobstant des délais abusifs, toutefois, rappelons que la pauvreté touche un enfant sur 5 et que si la monoparentalité est une prévalence, ces mesures devraient concerner l'ensemble des ménages modestes où les femmes sont contraintes de temps partiel et où la précarité progresse de plus la politique d'austérité à dégrader les services de la CNAF, soumis à des restitutions d'effectifs alors qu'elle devrait assumer alors qu'elle devait assumer les réformes de l'APL et le traitement des dossiers multiplie les retards ces situations dégradées ont à voir avec un partage des richesses, de plus en plus inégalitaire qui prive notre protection sociale des moyens de relever les défis du vieillissement et de la prévention un PLFSS qui apporte quelques mesures bienvenue mais perpétue une gestion comptable sans réflexion critique sur sa partie recettes, nous appelons un changement de paradigme d'autant que pour l'hôpital public, les professionnels alerte, ça se dégrade et ça se dégrade très vite et que nous approchons du moment de bascule ou l'effondrement du système de santé sera notre lègue à la nouvelle génération, chers collègues, mais le groupe écologiste restera donc merci, je vous remercie. La parole est maintenant Monsieur Abdallah Hassani pour le groupe RDPI pour 4 minutes. Monsieur le président. Mesdames, messieurs les Ministres, madame la présidente de la commission, affaires sociales et Madame la rapporteure générale les l'examen du PLF était moment d'importance, il est pour l'accès aux soins et la protection de nos. Concitoyens pour le soutien aux familles face à la précarité pour l'avenir de nos enfants, il est. Oh non, professionnels de santé, dont je tiens ici à saluer le dévouement et pour la région. Médical cette année, le Sénat a un rôle particulier, nous aurons à débattre des sujets centraux qui pour certains n'ont pas encore été discutés dans un hémicycle en profondeur, je pense à la prévention, aux mesures de soutien pour les familles monoparentales à l'organisation des soins sur notre territoire, ce texte est un engagement fort du gouvernement,

elle permettra la prise en charge. Deux 3 rendez-vous de prévention aux âges. Clés pour protéger nos concitoyens ou diagonales diagnostiquer un amont certaines pathologies, c'est avec une même ambition que nous avions souhaité avec l'autre groupe RDPI un amendement a déclaré hélas qui recevable visant à expérimenter. La prise en charge d'une consultation lors de l'adolescence, destiné à prévenir les troubles mentaux, il nous faudra. être attentif à cette problématique, des mesures ont été initiés comme la prise en charge des rendez-vous en psychologie votée l'an passé, nous croyons fondamental d'assurer toutefois une prise en charge plus amples, des troubles mentaux qui pour près de moitié, c'est leur l'OMS sont présents dès 14 ans, pour ce qui concerne mon département Mayotte je salue l'effort pour l'effort fait pour accélérer la convergence sociale, l'article trente-huit étant enfin à Mayotte la complémentaire santé à des conditions de revenus adapté au faible niveau de vie de ses habitants, du chemin reste à faire certaines prestations sont encore inexistantes à Mayotte ou servi avec des montants inférieurs et des conditions plus restrictives, l'article sept qu'un Sécurise par ailleurs l'exonération de la contribution spécifique d'assurance maladie applicable à Mayotte, ces 2 articles montrent que l'État, hé bien, à côté des Mahorais en tout cas c'est notre sentiment, faire que les territoires ultramarins demeure au coeur des innovations public nous proposerons qu'un territoire ultramarin soit sélectionné dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 24 qui vise à améliorer l'accès aux soins sur les territoires sous-dotés, il est un autre nécessaire de s'interroger sur les causes de la prévalence très élevé de l'obésité dans ces territoires, c'est un vrai problème de santé publique, un rapport publié en juin par mes collègues des Affaires sociales a souligné la spécificité des enjeux ultra- marins, le projet de loi présenté aujourd'hui porte des mesures d'encadrement et de contrôle nécessaires tant pour prendre en compte les pratiques nouvelles que pour agir face à des situations d'abus, il contient des expérimentations visant à faciliter et harmoniser le parcours de soins tout en intégrant une responsabilité collective pour assurer la permanence des soins. Nous avons souhaité porter sur ce sujet. Difficile, plusieurs amendements avec une attention particulière sur les zones les moins dotés, comme vous le constatez ce texte porte à la fois des engagements financiers fort et des avancées concrètes pour chaque Français, c'est pourquoi le groupe des pays votera ce texte. Merci, merci, cher collègue là. Parole et maintenant Monsieur. Bernard Jomier pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour sept minutes.

monsieur le président, Mesdames et messieurs les ministres, madame la présidente, madame la rapporteure, mes chers collègues. Tout d'abord, ce texte qui est issu du 49 3 un avenir incertain, comme je le disais tout à l'heure et le gouvernement aurait pu d'ailleurs saisir le fait qu'il était né du 49 3 pour nous proposer un projet de loi structuré et cohérent, or il hésite encore une fois, entre une loi de finances et une loi d'organisation du système de santé loi par ailleurs que nous appelons Monsieur le Ministre de nos voeux et c'est indispensable car, par ailleurs, depuis la crise sanitaire, les collectivités territoriales se saisisse de l'organisation du système de soins dans les territoires. Contribuant ainsi à modifier la gouvernance en santé du pays, hé oui, il nous faut partir des besoins des territoires pour ensuite céder aux arbitrages budgétaires, l'outil de régulation qui est l'Ondam montre ses limites, la maîtrise qu'il porte s'impose avant toute délibération sur les besoins en matière de santé dans nos territoires comme au Parlement, où aucun débat sur les besoins sociaux de la nation n'a lieu en amont de la délibération budgétaire pourtant passer d'une logique d'offre à une logique de besoins en santé est primordiale, mais dans ce texte, vous en restez à la politique de l'offre, l'an dernier, nous regrettons un budget de fin de quinquennat sans grande nouveauté cette année, nous espérions un budget de la Sécurité sociale à la hauteur d'un président de la République réélu mais le souffle est court, le gouvernement revendique d'inscrire ce budget dans la continuité de ce de 2010 à 2000 19 ans trajectoire de réduction des déficits, cette mise à l'équilibre s'était faite au détriment de l'hôpital public, à l'époque, ce choix était déjà discutable, aujourd'hui il n'est pas supportable l'Ondam hors dépenses de crise évolue de 3,7 une évolution qui est nettement inférieur à l'inflation actuellement de plus de 6 % et probablement entre 4 et 5 l'an prochain en définitive : malgré une communication volontariste du gouvernement ce budget post-Covid réduit les moyens financiers attribués au système de soins. Par ailleurs, nous affirmons avec force que les comptes de la Sécurité sociale pourraient être en équilibre, en témoigne l'augmentation depuis 2017 des exonérations de cotisations sociales en 2018, elles représentaient moins de 40 milliards d'euros, contre 60 et 11 milliards en 2023, bien que des baisses de cotisations sur les bas salaires puissent être utile, la majorité d'entre elles relèvent d'une politique fiscale favorisant les plus aisés, le Conseil d'Analyse économique publiée en 2019 une note intitulée baisses de charges Stop ou encore est-il recommandé l'abandon des exonérations de cotisations sur les salaires supérieurs à 2 5 SMIC au motif qu'elles sont sans effet sur l'emploi, j'ajouterai que le gouvernement a décidé de faire porter le coup du Covid à la sécurité sociale, ce qui représente cette année une perte de recettes de 17,7 milliards d'euros, alors qu'il serait plus pertinent que l'État prenne en charge cette dette et donc, si l'on prend en compte ces sommes non seulement les administrations de Sécurité sociale dégagerait un fort excédent, mais de même elle nous permettrait d'accroître les investissements nécessaires au système de santé de façon plus globale nous désapprouvons cette logique politique de fléchage de la dépense publique vers des exonérations et des allégements de charges, car notre pays a besoin d'investissements structurels stratégique et de long terme, la dépense publique dans notre pays est passée en 40 ans de 46 à 55 % du PIB certes. Mais il faut aller au bout de l'analyse car un tiers seulement et consacrée au fonctionnement de l'État et ses services, c'est-à-dire payer les agents payer les achats, les prestations pour la santé, pour la justice, ou pour l'école, 2 tiers de la dépense publique, ce sont maintenant des transferts aux ménages et aux entreprises, et donc à la lecture de ces chiffres, on comprend ce qui paraît paradoxal à beaucoup de Français c'est-à-dire qu'alors que la dépense publique augmente c'est la décrépitude de nos services publics, hé bien en 2020 nous ne consacrons pas plus d'argent à nos services publics qu'à la fin du septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Par contre, en seulement 5 années de 2018 à 2023, les exonérations de cotisations sont passées de 39 à 71 milliards d'euros, c'est votre choix, c'est votre politique et elle détruit nos services publics, dans celui de la santé concernant la branche maladie, vous connaissez évidemment Monsieur le Ministre, la gravité de la situation dans laquelle se trouve notre système de soins, vous connaissez nos hôpitaux publics qui sont en voie d'affaissement d'effondrement, diront certains, et pourtant ce budget de la Sécurité sociale qui devait apporter des réponses structurelles après la crise du Covid et ce qu'il ce sujet majeur, l'hôpital est le grand absent de ce budget car vous continuez mesdames et messieurs les Ministres, a argué des revalorisations, certes bienvenue du Ségur de la santé pour illustrer votre investissement à l'hôpital mais c'est largement insuffisant et preuve en est les ajouts ces dernières semaines de montant supplémentaire bienvenu, mais qui traduisent un pilotage à la petite semaine et nous assistons à l'hémorragie de personnel et les soignants quittent l'hôpital et des services d'urgence doivent être réduits, parfois même fermé la direction statistique de vos ministères l'adresse, indique que les capacités hospitalières ont subi des contraintes de personnel ne permettant pas de maintenir les lits, la réalité de ce budget, c'est ce que ce seront des personnels en moins, c'est que ce sont des services qui ferme le tiers parfois la moitié de leur dit ce sont des activités de soins qui partent vers le privé, ce sont des patients qui sont trimballées d'une région à une autre et pour ce qui est des soins de ville, la dépense augmente de seulement 2,7 % soit moitié moins que l'inflation votre majorité désorganise le parcours de soins texte après texte Maxime si vous Monsieur le Ministre, contrairement à votre prédécesseur, nous prenons acte de votre volonté de renvoyer à la négociation un certain nombre de questions sur la prévention. Un texte ne peut se révéler revendiqué ambitions en matière de prévention quand elle traite de la sorte, le tabac et l'alcool, car cette mise en place d'une campagne de taxation programmée du tabac là la campagne pardon sous les gouvernements précédents, a permis de réduire le tabagisme dans notre pays, mais en ce début de quinquennat le gouvernement s'est contenté d'aligner le tabac sur l'inflation, et pire, vous avez reculé sur le tabac, chauffé, suite à la présence du ministre des Comptes publics au congrès des buralistes, on comprend où se fait la santé publique sur l'alcool, il n'y a simplement rien dans ce budget, vous l'avez compris, nous ne pouvons pas nous satisfaire de ce budget imposée en cette période charnière des économies au système de soins est irréaliste et dangereux, le 1er, texte de ce gouvernement qui concerne la santé et peu ambitieux et mal financée, nous proposerons de re-certifier sa trajectoire pour mettre en oeuvre les réformes nécessaires pour que notre sécurité sociale, assure à l'avenir, l'ensemble des missions de protection sociale dans notre démocratie peut être fier, je vous remercie.

Monsieur le président, messieurs et Mesdames les Ministres, mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, monsieur le ministre de la Santé en 6 ans votre politique de santé n'a ni amélioré les conditions de travail du personnel, ni même le sort de nos concitoyens, bien au contraire, alors oui, me direz-vous, il y a eu la crise du Covid et ses conséquences, mais vous avez préféré faire payer au budget de la Sécurité sociale, les dépenses liées à la crise, alors que celle-ci aurait dû être imputés sur le budget de l'État, nous vous proposons à travers plusieurs amendements, enfin pour ceux qui ont survécu aux articles 40 45 et j'en passe car c'est l'hécatombe de changer de braquet, ces amendements ont été rédigés au contact des personnels de santé du médico-social des associations, des citoyens, ils ne sont pas dogmatique, mais permet une politique qui rompt avec votre logique libérale qui n'a pas fait ses preuves, lorsque quelque chose ne fonctionne pas et votre politique de santé n'a pas fait ses preuves, on change de méthode, on essaie d'améliorer, d'écouter, de prendre en considération les remarques, on n'a jamais raison seul, alors vous avez encore si vous le souhaitez, l'occasion avec ce Plfss 2023 de revoir votre copie partout dans le pays, notre système de soins craque les soignants manquent à l'appel, ils sont fatigués de ne pèse 30, tendu, nos concitoyens ont de plus en plus de mal à trouver un médecin de ville, même en cas d'urgence, pour rappel, 6 millions de Français n'ont actuellement plus de médecin traitant les maires, les élus sont nombreux à tirer la sonnette d'alarme pour leur population en urbain ou en ruralité nous vous proposons donc de pour pallier à l'urgence d'augmenter les moyens des territoires, des hôpitaux, cela passe évidemment par un budget ambitieux, une des seules alternatives que vous nous proposez dans une course de vitesse avec la droite sénatoriale, d'ajouter une année supplémentaire aux études de médecine, celle-ci passant de 9 à 10 ans cette mesure s'est fait sans concertation, de plus elle incite incite les internes en 9ème année à aller dans les déserts médicaux à moindres coûts, encadrés par un médecin senior mais savez-vous que la plupart des territoires manque cruellement de médecins seniors pour encadrer ces internes : pensez-vous réellement régler le problème de cette façon, le comble c'est qu'avec cette mesure, d'une année supplémentaire vous entraîner une année blanche pour l'installation de nouveaux médecins en faisant cela vous aggravé la situation, à l'inverse, nous vous proposons d'augmenter les moyens des universités pour former davantage de médecins chaque année l'Ondam est lui aussi sous-évalué, fixé à 3 7 % quand l'évolution naturelle des dépenses de santé est établi à 4 % par la commission des comptes de la Sécurité sociale, soit, soit 0,3 point de moins et si l'on compare cet Ondam à l'inflation qui est de 6 2, le compte n'y est pas au total ce sont un virgule 7 milliards d'euros qui disparaissent de la santé, c'est donc un budget au rabais que vous nous présentez aujourd'hui un budget décevant, qui n'est pas à la hauteur des besoins, ce manque d'ambition se traduit également sur le plan de l'autonomie, vous mettez en avant le recrutement de 3000 infirmiers, aides-soignantes dans les EPHAD ce qui est largement insuffisant par rapport aux besoins estimés, notamment pour atteindre un encadrement d'un personnel un résident, 170 millions d'euros pour recruter dans les EPHAD représente à demi-poste de plus de 7000 pas de France, alors que les besoins sont estimés à 300000 ce premier Plfss depuis la publication du livre de Victor Castanet les fossoyeurs, sur la gestion calamiteuse des Ephad et là aussi décevant, le renforcement des pouvoirs d'inspection de l'Inspection générale des affaires sociales n'à ce titre, pas suffisant et nous demandons le remboursement automatique des subventions publiques indument perçues par Orpea malheureusement vous avez jeté aux orties la loi grand âge autonomie pourtant promise il y a quelques mois par votre gouvernement dans son rapport annuel sur le financement de la Sécurité sociale, la Cour des comptes dénonce l'étatisation de la Sécurité sociale via le remplacement croissant des cotisations par l'impôt de 90 % à la fin des années 1980 la part de ses revenus issus du travail est tombé à 50 pour 100 depuis 2019, le système de tuyauterie entre le budget de l'État et la sécurité sociale est devenue tellement multiple et complexe que la Cour des comptes appelle elles-mêmes à y mettre fin, dans la même veine, des tours de passe-passe, le gouvernement a inscrit dans ce projet de loi, le transfert précipité du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco vers l'Urssaf, alors que le 21 juin 2022, le rapport de la Mecque sur l'unification du recouvrement social que nous avons fait avec mon collègue René-Paul Savary avec lequel je n'ai donc pas que des désaccords préconisé de reporter ce transfert les difficultés techniques de ce transfert et les risques pour les assurés, d'une perte de contrôle sur leurs cotisations retraite justifie l'abandon de ce projet, d'ailleurs, l'ensemble des organisations syndicales et patronales y sont opposés, écoutons-les, mais le gouvernement n'en tient pas compte et accélère à l'article 6 le transfert du recouvrement des 87 milliards d'euros de cotisations Agirc-Arrco de même sur les retraites, si le gouvernement a finalement reculé, c'est pour mieux sauter la réforme promise divise tellement que même vos alliés ont renâclé devant l'obstacle, récusant la volonté de passage en force, qui est votre marque de fabrique la précipitation et la détermination affichée du président et de son gouvernement sont pourtant à contre-courant des perspectives du conseil d'orientation des retraites dont le dernier rapport démontre que les dépenses de retraite du pays resteront stables dans le temps à 13,9 % du PIB et que si les régimes de pensions deviennent légèrement déficitaire de 2022 à 2032, c'est essentiellement parce que l'État prévoit d'économiser sur la masse salariale publique en redisant les traitements des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, comme chaque année, nous aurons le débat sur l'allongement de l'âge légal de la retraite au Sénat avec l'amendement du rapporteur de la branche vieillesse, René-Paul Savary, qui prévoit le report près groupe progressif de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, notre groupe porte à l'opposé, l'abaissement de l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans ce PLFSS 2023 1er budget de la nation va encore aggraver les inégalités, il ne sera pas ce que vous annonciez dans le journal Le Point, celui de la santé et de la solidarité, celui qui vous rendez si fier, il n'en sera rien puisque vous avez décidé de façon autoritaire d'actionner le 49 3 alors que ce budget de la Sécurité sociale, aurait dû être l'occasion d'un débat constructif avec l'ensemble des partenaires, la balle était dans votre camp, vous n'avez pas su la saisir, vous avez préféré passer en force, nous voterons contre ce PLFSS 2023. Merci, cher collègue. La parole est maintenant monsieur Jean-Marie Vanlerenberghe pour le groupe Union centriste pour sept minutes. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les Ministres, madame la rapporteure générale chère Élisabeth, madame la présidente, c'est-à-dire Catherine mesdames messieurs les rapporteurs, chers collègues de partout monte la même complainte : il faut plus, plus d'argent pour l'hôpital, plus de médecins et de soignants, plus de crèches, plus d'argent pour les retraites : plus de moyens pour la 5ème, branche dont vous parlera d'ailleurs Jacques Jocelyne Guidez, bref autant de questions, mesdames et messieurs les Ministres, pour le gouvernement et pour nous, une seule question : le PLFSS 2023 y'répond-il vraiment. En apparence, je dirais oui. Avec 601 milliards pour les 5 branches des dépenses sont supérieurs de plus de 12 milliards à la prévision et le déficit total est néanmoins ramené à 6 milliards 8 contre 17 8 l'an dernier l'Ondam progresse de 3 7 % hors crise Covid donc à Champ constant, ce qui est significatif, mais les apparences ne sont-elles pas trompeuse, seules 2 branches sont à l'équilibre, la famille, la TMP et les hypothèses ne sont-elles pas trop optimiste, l'assurance maladie accuse encore un déficit de 6 mias 6 milliards et demi et l'hôpital va de crise en crise urgences pédiatrie psychiatrie et ce n'est pas en ponctionnant 2 milliards à la branche famille qu'on sauvera l'hôpital. L'hôpital est malade, mais c'est tout notre système de santé qu'il faut soigner, il est à bout de souffle son mode de fonctionnement est à revoir, Emmanuel Macron a promis de ramener la tarification à l'acte à 50 % % pour mieux rémunérer la qualité et le travail en équipe, nous nous attendons donc Monsieur le Ministre, un plan d'action et surtout des actes pour apporter à l'hôpital un financement sain et pérenne, le mode de gouvernance aussi est à revoir, et point n'est besoin d'une loi supplémentaire, nous avons vu que les établissements, ils sont parvenus le CH de Valenciennes en particulier expérimente un mode de fonctionnement anti-pyramidal anti-bureaucratique et ça marche plus d'autonomie, plus de délégation, on fait confiance aux médecins et à leurs équipes pour raccourcir les décisions au bénéfice bien sûr des patients et du budget qui ne consacre plus que 5 % à l'administratif contre 5 fois plus ailleurs le directeur canalise les énergies quilibre le budget et entretien effectivement la paix sociale, monsieur le Ministre, la solution est là, n'attendons pas pour la généraliser, il faut aussi, vous le savez, fluidifier le système de soins pour désengorger l'hôpital et ses urgences la clé existe L C Pts la coordination ville hôpital est essentielle pour lutter contre les déserts médicaux et quand je dis hôpital je pense bien sûr aussi aux établissements privés, l'amélioration de la permanence des soins et l'accès aux soins passe en effet par la mise en place partout des ces BTS, comment accepter que 40 % des médecins de ville seulement assure la garde de nuit et le week-end, si les médecins veulent retrouver du temps médical il doit déléguer aux autres soignants une partie de leur travail, je salue d'ailleurs l'accord conclu en ce sens entre les différents ordres Monsieur le Ministre, vous parlez souvent de votre boîte à outils, les solutions existent et elle marche, il faut les diffuser les élus locaux sont prêts à faire les efforts nécessaires pour que l'égalité qui est inscrite au fronton des mairies s'applique aussi dans l'accès aux soins, mais une question se pose, c'est l'économie du système, les professionnels réclament des plans pluriannuels pour anticiper des évolutions thérapeutiques et permettre à notre pays de rester à la pointe du progrès dans ce domaine, cela mérite une très grande attention et la dernière question concerne les ressources, la première piste tous les ministres ont utilisé, c'est celle des économies, la source n'est pas tari, elle est même je crois abondante, mais encore faut-il ne pas se tromper, longtemps, longtemps, la ressource humaine a été pressurés mal rémunérés le Ségur à apporter un effet salvateur, mais elle doit être poursuivie et cela coûte d'autres pistes sont donc à privilégier les actes redondants et inutiles représentent 20 à 30 % de notre système de soins, soit 40 à 60 milliards de dépenses à revisiter la HAS s'y emploie, mais vous avez ciblé, à peine plus d'un milliard d'économies sur la radiologie, la biologie, les médicaments dans votre projet, c'est bien mais insuffisant par ailleurs un autre demande l'estimation des fraudes aux cotisations et aux prestations est en cours, la CNAB bons élèves ont rendu leur résultat par contre la CNAM est très en retard, si nous voulons éviter l'exploitation fantasmée du montant de ces fraudes, il faut des chiffres et rapidement, enfin un mot sur les retraites, le déficit et la dette se creuse une réforme s'impose, mais attention, si nous ne voulons pas mettre des millions de personnes dans la rue, il faut qu'elle soit comprise et acceptée l'amendement que notre collègue René-Paul Savary, dont je salue la compétence et la constance aussi dans l'effort il répond-il partiellement seulement à mes yeux, en effet, si je crois utile la réunion d'une convention nationale pour préparer la loi parce que je suis partisan du paritarisme par contre je ne partage pas le recul à 64 ans de l'âge de départ dit et ce qu'on dit, le président de la République et la première ministre 64 ou soit ça 5 ans ne sont pas des totems à titre personnel, je serais plutôt partisan d'une fenêtre de départ comme le préconise, économiste, Jean Tirole et Olivier Blanchard, dans leur rapport de 2021, l'âge moyen de départ étant d'ailleurs de de 62 ans et demi on pourrait simplement le reculé à 63 ans.

le relèvement des petites pensions l'insertion des chômeurs de longue durée et par justice j'entends aussi le maintien au travail des seniors licenciés prématurément selon Jean Hervé Lorenzi, l'activité des seniors pourraient se de plus rapporter 13 milliards en disant

Merci, cher collègue. La parole est maintenant Madame Esther Benbassa pour les non inscrits pour 3 minutes. Monsieur le président, mesdames les rapporteurs, monsieur le ministre, mesdames les ministres, mes chers collègues ce PLFSS que vous souhaitez imposer coûte que coûte, manque d'ambition et de sincérité, nous sortons à peine de la crise sanitaire et vous nous promettiez après le Ségur de la santé que le personnel soignant serait écoutez que le l'hôpital public connaîtrait une véritable restructuration que l'ensemble des Français aurait enfin un système de santé digne de ce nom, il est vrai aussi que tant d'années de négligence et de casse ne se rattrape pas d'un coup de baguette magique, nous attendions un projet de loi de financement de la Sécurité sociale, plus fort, plus ambitieux, laissant plus de place à la justice sociale, il y avait un effet de quoi faire le bilan du précédent mandat parle de lui-même, plus de 21000 fermetures de lits, fin 2019 la dette de l'hôpital public s'élevait à plus de 30 milliards des hôpitaux en faillite qui ferme des services d'urgence et de maternité et un personnel soignant complètement découragés et démissionnaire, pourquoi ce texte n'aborde-t-il pas les sujets qui fâchent, je pense notamment à la pénurie de main-d'oeuvre que connaît actuellement l'hôpital aux personnes âgées en perte d'autonomie aux Français des DOM-TOM, qu'on oublie trop souvent, enfin aux assistantes maternelles qui soit disant gagneraient 3 SMIC et qui pourtant vivent dans des conditions précaires, vous aviez aussi la possibilité de concrétiser la promesse du président de la République qui consistait à mettre la cause des femmes au coeur de sa politique, qu'en est-il réellement de la gratuité des protections hygiéniques pour toute de la lutte contre l'endométriose et de l'inégalité territoriale d'accès aux établissements de santé pratiquant l'IVG, enfin je ne souhaite pas allonger la liste mais ce projet de loi n'est pas une réponse sérieuse et convaincante aux enjeux colossaux de notre système de santé, j'ai une pensée pour mes collègues députés, qui ont travaillé pendant des jours pour amender ce projet de loi et qui ont vu leurs efforts réduits à néant la semaine dernière, bien que le 49 3 un outil constitutionnel, vous ne pouvez pas à ce point mépriser le travail parlementaire la menace, la menace du 49 3 ne plane pas au-dessus de nos têtes, certes nous mèneront les discussions jusqu'au bout pour améliorer votre copie, je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est maintenant Madame Véronique Guillotin, pour le groupe RDSE pour six minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame la présidente de la commission, mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues, je tiens d'abord à remercier la présidente de commission et nos rapporteurs qui nous ont permis d'entamer ses débats avec clarté et c'était pas simple la crise Covid s'éloigne mais gardons en tête qu'elle a été et qu'elle reste un marqueur fort de ce Plfss en ayant aggravé de manière inédite, nos comptes sociaux nos finances se sont toutefois redressé de manière spectaculaire, plus vite et plus fort que prévu, pour autant, selon les prévisions du gouvernement, le budget ne sera pas encore à l'équilibre l'an prochain et devrait se dégrader dans les années à venir, malgré des prévisions de recettes qualifiées d'optimistes par le Haut Conseil des finances publiques dans son avis sur le budget 2023 en même temps, les dépenses de santé paraissent sensiblement sous-estimé, notamment l'Ondam de ville avec 0 5 point de plus que le rythme d'avant Covid dans un monde à faible inflation et sans compter sur le virage ambulatoire qu'il faut poursuivre, voire accélérer quant au secteur hospitalier, la hausse de 4 virgule un pour 100, saluée par les acteurs du secteur questionne tout de même ces mêmes acteurs au regard de l'inflation de la hausse des salaires, du coût de l'énergie et d'une activité pas encore revenue à la normale, d'où la demande légitime pour certains hôpitaux de la poursuite de la garantie de financement, je reconnais la difficulté de l'exercice qui consiste à concilier à la fois la maîtrise de nos comptes sociaux, tout en répondant aux besoins de la population et au système de santé à bout de souffle, tout cela dans un contexte économique et social, plein d'incertitudes, malgré des efforts financiers importants consentis par le gouvernement, il faut le dire, malgré la 2ème place de la France dans les pays de la zone Euro qui consacrent la plus grande part de leur PIB à la santé, malgré sa 7ème place dans les pays qui consacrent pour la santé, le plus d'argent par habitant, le système notre système de santé est au bord de la rupture et force de constater que le dispositif législatif qui est le PLFSS j'ai mis quelques années à m'en rende compte, n'est pas vraiment adapté au pilotage de la transformation d'une politique de santé qui nécessite une vision de long terme cette transformation en profondeur ne peut me semble-t-il s'envisager qu'au travers une loi de programmation et d'orientation et de programmation pluriannuelle qui fixerait un cap tout cela accompagné d'une étape de décentralisation sur des sujets tels que la prévention, l'éducation de la santé, mais aussi des réformes structurelles, je pense à l'art, forme des retraites à la loi, grand âge et un financement de la Sécurité sociale plus efficient et plus lisible mais disons-nous aussi que la problématique centrale et le manque de médecins, et que l'on ne peut l'imputer à ce gouvernement avec les remarques que je viens de faire j'en reviens au PLFSS et à ces mesures concrètes dont nous avons à débattre et notamment à la question de l'accès aux soins, qui me paraît central, il prévoit un meilleur partage des tâches pour libérer du temps aux médecins et valoriser les professionnels de santé non médicaux, notre groupe est favorable aux diverses mesures d'extension d'autorisation de vaccination favorable à permettre aux infirmières de signer des certificats de décès à l'expérimentation d'accès Direct pour les IPA nos amendements visait à accélérer le déploiement de ces mesures, elles ont malheureusement été frappée d'irrecevabilité, nous le regrettons, car le temps presse et nous souhaitions accélérer ce mouvement, compte tenu du nombre important de médecins qui atteindront l'âge de départ à la retraite dans les années à venir, nous sommes favorables à faciliter le cumul emploi-retraite, les incitant ainsi à poursuivre leur activité, la simplification des démarches administratives via le guichet unique, tout comme la régulation de l'intérim, vont dans le bon sens, l'autre grand sujet, celui de la prévention, cela a été dit, c'est la première fois que nous avons un ministre de la Santé et de la prévention et quand on sait à quel point la prévention et le soin sont liés, le sujet n'est pas anodin, sans cynisme, il revêt aussi un caractère d'importance pour nos finances publiques prévenir coûte effectivement moins cher que guérir ce Plfss prévoit aussi plusieurs rendez-vous de prévention remboursé par la Sécurité sociale, à des périodes clés de la vie afin de repérer et traiter les fragilités liées à l'âge où les addictions tout en promouvant l'activité physique et un mode de vie sain, laissons les professionnels organisés de manière la plus efficace possible ces journées de prévention, nous voterons bien sûr cette mesure, tout comme celles qui permettent un meilleur accès au dépistage des infections sexuellement transmissibles et à la pilule du lendemain, j'en viens enfin la mesure qui occupe une bonne partie de nos débats depuis plusieurs semaines maintenant, la réforme du 3ème cycle des études médicales cette année professionnalisante est utile pour bien préparer les jeunes médecins à leur futur exercice ambulatoire si elle répond à leurs besoins par un encadrement et un contenu pédagogique adapté, alors je n'ai aucun doute qu'ils seront nombreux à s'installer là où ils ont été bien accueillis et bien formées, mais la communication et la rédaction de cet article dévoile le véritable objectif poursuivi par certains, lutter contre la désertification médicale en déployant un bataillon de jeunes en formation, je crois, les déclarations de nos ministres sincère quand il se positionne en défaveur de la coercition, alors pourquoi ne pas clarifié nos intentions en mettant la formation au coeur de la réforme est au coeur de la rédaction de cet article, je proposerai ainsi d'amender l'article sur 3 critères qui me paraissent essentiels : tout d'abord la supervision doit être effectuée par un maître de stage des universités cette année supplémentaire doit pouvoir être réalisés sur tout le territoire, en effet, la limitation zone sous-dense dans la définition et d'ailleurs trop imparfaite puisqu'elle concerne 80 % du territoire est une mesure à la fois inefficace voire contreproductive en période, je précise, de pénurie de médecins, enfin, autorisant la liberté d'opter pour un stage en hôpital de proximité, en complément du stage ambulatoire qui répond tout autant aux besoins des territoires au décloisonnement ville hôpital que nous appelons de nos voeux et aux aspirations des nouvelles générations pour l'exercice mixte pour le reste, nous aurons l'occasion mes collègues du groupe RDSE et moi-même, de défendre nos amendements et de nous prononcer sur les autres mesures au cours de cette semaine de débats, je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est maintenant à Madame Florence Lasserre pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes. Mesdames et monsieur le ministre, monsieur le président, mes chers collègues, nous allons examiner le premier projet de loi de financement de la législature, je commencerai par évoquer quelques chiffres ce projet de loi porte sur près de 600 milliards d'euros de prélèvements obligatoires et de dépenses publiques, il prévoit une diminution forte du déficit de la Sécurité sociale, qui passera à 7 milliards d'euros, contre 18 milliards en 2022, tout en se fondant sur une croissance économique très optimiste de 1 % en France, là où les instituts prévoient 0 6 % les déficits sont inquiétants et vos hypothèses budgétaires trop optimistes concernant l'accès aux soins à l'hôpital et le grand oublié de ce PLFSS j'aimerais évoquer la situation particulière de la pédiatrie et de la santé des jeunes en premier le je souhaite attirer votre attention sur un phénomène inquiétant dans une étude publiée en mars 2002 dans cette des chercheurs de l'INSERM ont constaté une hausse de décès de nourrissons entre 2000 19 ces travaux indiquent une augmentation de la mortalité infantile de 7 % alors que la France figurer parmi les meilleurs élèves, elle a chuté de la 7ème à la 25ème place entre 1989 et 2017 or, malgré ces chiffres inquiétants : la réduction du taux de mortalité infantile n'est actuellement pas considéré comme une priorité de santé publique depuis début octobre, les urgences et services de réanimations pédiatriques des hôpitaux de tout le pays sont saturés du fait d'une épidémie de bronchiolite des plans des plans blancs sont déclenchés, mais cela conduit une fine et à déstabiliser un peu plus notre système hospitalier : comment en est-on arrivé là les capacités d'accueil des services se dégrade en région du en raison du manque de personnel soignant qui a abouti à la fermeture de 15 à 20 % du lit, face à la dégradation de la situation, vous avez annoncé, dans un 1er temps le déblocage d'une enveloppe de 150 millions d'euros à partager entre les services en tension, mercredi dernier, c'est une enveloppe de 400 millions d'euros que vous annonciez en répondant à la crise de la pédiatrie ces mesures non structurante. Ne permettront pas la survie de la pédiatrie et l'arrêt de la dégradation des soins aujourd'hui 44 % des pédiatres libéraux ont plus de 60 ans la répartition sur le territoire est inégal 8 départements comptent même moins d'un pédiatre pour 100000 habitants dans ce contexte, les médecins généralistes sont appelés à jouer un rôle croissant mais ils demeurent inégalement formés à la médecine de l'enfant, l'article 20 du PLFSS étant la compétence de l'administration de prescription des vaccins par les pharmaciens, sages-femmes, infirmiers, des délégations de tâches oui mais pas n'importe comment, il ne faut pas d'déconnecté la vaccination du suivi médical et de l'examen obligatoire des enfants, l'accès au pédiatre en 1er recours dans le parcours de soins ambulatoires pour tous les enfants doit être maintenu, les puéricultrices et auxiliaires de puériculture doivent voir leurs compétences valoriser la pédopsychiatrie également manque cruellement de moyens, alors que les confinements la distanciation sociale le port du masque, né de la crise sanitaire provoque des effets majeurs sur la santé mentale des jeunes, idem pour le secteur de la psychiatrie, qui est complètement sinistrée, auquel le gouvernement n'apporte aucune mesure de soutien, la situation de l'hôpital public appelle des efforts courageux et des réformes structurelles, les professionnels de santé attendent des mesures fortes, notamment en terme d'organisation, de gestion et de répartition plus juste des moyens ce PLFSS propose l'interdiction de l'intérim médical, notamment pour les jeunes diplômés, médecins ou infirmiers c'est souhaitable, mais l'intérim des jeunes diplômés, n'est pas le seul à fragiliser le fonctionnement des établissements de santé, la qualité, la continuité des soins, la commission des affaires sociales a renforcé les dispositions inscrite dans le texte, en indiquant que l'intérim ne pouvait pas être le seul mode d'exercice à plein temps des professionnels de santé, je proposerai personnellement un amendement pour limiter la période d'intérim à cinq ans, dans le service public hospitalier, l'article 22 qui prétend rénover la vie conventionnelle ne modifie en réalité qu'à la marge les règles encadrant les conventions conclues entre les organisations représentatives des professions de santé, l'assurance maladie, la mesure la plus discutable et sans doute l'ajout parmi les thèmes pouvant être abordé à l'occasion de négociations pour la plupart des professions du conventionnement conditionnel ma conviction en tant que médecin et que ce type de mesure ne sert pas à grand chose, dans un contexte de pénurie médicale généralisée, près de 90 % de du territoire manque de médecins libéraux, l'exaspération monte chez les machins et les étudiants vous réponse reste insuffisant pour faire face à la paupérisation du secteur médical, les établissements de santé nous alertent sur leurs charges et libéraux attendent des revalide réalisation et le secteur du médicament, ce plan d'économies drastiques des réponses doivent être apportées rapidement à ces problèmes avec des mesures structurelles et pérenne, nous souhaitons notamment une augmentation du nombre de places pour les étudiants en médecine, un redoublement possible de la première année, une tarification des actes fortement revalorisé pour tous les modes, exercice hospitalier comme libéral, je vous remercie de votre attention. Merci, cher collègue. La parole est maintenant à monsieur Xavier Iacovelli pour le groupe RDPI pour cinq minutes. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les Ministres, madame la rapporteure générale, madame la présidente, chers collègues, avec un déficit de 17 8 milliards d'euros en 2022, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2023 tablent sur un déficit de 6 8 milliards si cette perspective est encourageant je souhaiterais ici rappeler les enjeux auxquels nous sommes confrontés, ce projet de loi de financement de répondre un double objectif : tout d'abord celui de réduire les déficits budgétaires tout en pas ça en s'attaquant aux problématiques que vivent nos concitoyens en matière de santé au quotidien mais il doit également poser les fondations d'un système plus ambitieux et plus juste qui protège tous les Français, c'est cette vision que notre groupe ont emporté avec une politique sociale forte est synonyme de progrès en se projetant à l'avenir et à l'horizon 2025 ce PLFSS pose les fondations dans notre pays a besoin afin de préserver et d'améliorer notre système de santé et de protection sociale, je pense tout d'abord à des mesures volontaristes en matière de prévention et d'accès aux soins avec la mise en place du rendez-vous de prévention aux âges clés de la vie, je pense au dépistage sans ordonnance des infections sexuellement transmissibles, sur le modèle du dépistage du VIH ou encore à l'accès gratuit et sans ordonnance, pour toutes les femmes à la contraception d'urgence, alors même que seulement 10 % sont actuellement remboursés. Cette prise en charge doit, comme le prévoit le ce s'accompagner d'une information renforcée vis-à-vis de toutes les femmes et en particulier des plus jeunes d'entre elles il s'agit là de mesures en matière de santé des femmes dans la continuité de l'action du gouvernement et de la majorité présidentielle depuis 2017 et je pense notamment à la gratuité de la contraception pour toutes les femmes de moins de 25 ans, il me semble par ailleurs essentiel d'entamer une réflexion sur la précarité menstruelle qui touche de nombreuses femmes et notamment les plus jeunes au moment où 13 % des étudiantes déclarent avoir dû, faute de moyens, choisir d'acheter entre protections périodiques ou produits de première nécessité, la lutte contre toutes les inégalités d'accès à la santé qui abîme notre pacte social doit être une priorité, il s'agit d'une mesure de justice sociale, à l'heure où près de 4 millions de Français vivent dans une zone sous-dotée en professionnels de santé, je pense notamment à la mise en place du guichet unique dans chaque département, qui vise à simplifier l'installation de nouveaux médecins ou encore à la création d'une 4ème année d'internat de médecine générale une année supplémentaire sera consacrée à des stages en cabinet médical, en particulier dans les zones médicalement tendu, il s'agit là aussi d'un signal fort qui pose les bases d'une politique visant à réduire les inégalités sur le territoire national, à la politique pour la politique familiale ce PLFSS se veut également ambitieux en matière de politique de la famille, je pense au complément de libre choix, de mode de garde le CMG qui doit être réformé, aujourd'hui les parents employant une assistante maternelle sont trop défavorisé par rapport aux familles qui recourent à la crèche, notre groupe se félicite donc des propositions avancées sur ce sujet avec le nouveau mode de calcul du CMG emplois Directs qui permettra de rendre l'accueil pour les assistantes maternelles aussi accessible que la crèche et d'harmoniser le reste à charge entre ces 2 modes d'accueil, d'autre part, les études montrent également que les enfants des familles monoparentales sont 2 fois plus touchés par la pauvreté, que les enfants que les autres enfants je tiens ici à saluer le renforcement des aides à destination des familles monoparentales notamment l'allocation de soutien familial destiné aux parents isolés, qui sera revalorisée de 50 c'est une bouffée d'oxygène pour ses parents et ses enfants qui font face à des situations problématiques enfin notre groupe se félicite du travail mené sur ce PLFSS 2023 qui pose les bases d'une politique plus juste et qui tend à améliorer notre système de santé pour les années à venir, nous proposerons détendre les rendez-vous de prévention au diagnostic précoce des troubles de santé mentale, celui-ci est essentiel pour assurer une bonne prise en charge de ces pathologies, alors que nous savons que la psychanalyse et la psychiatrie pardon constitue le 1er poste de dépenses de l'assurance maladie, loin devant le cancer et les maladies cardiovasculaires, nous entendrons également mener une réflexion sur les inégalités persistantes entre les femmes et les hommes en matière de contraception cette réflexion ne semble essentiel pour établir une meilleure répartition de la responsabilité de la vie sexuelle, alors que l'achat des moyens de contraception est majoritairement réalisés par les femmes. Pour toutes ces raisons, en complément des propos de mon collègue Abdallah Hassani, le groupe RDPI soutiendra pleinement les mesures et l'orientation de ce budget, un budget ambitieux qui répond au double objectif de réduction du déficit toujours et toujours plus de protection pour les Français, un budget de justice sociale qui finance des progrès nouveau et fait le choix de renforcer le volet prévention et notre système de santé un budget, enfin qui porte des réponses concrètes aux déficits structurels auxquels est confronté notre modèle social, de santé et qui devra nécessairement être modernisés, je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est maintenant Madame Michelle Meunier, pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour 4 minutes. Monsieur le président, Mesdames les Ministres Monsieur le Ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure générale, chers collègues, que pensent les sénatrices et sénateurs socialistes sur la branche autonomie si l'on s'en tient aux 4 articles présents dans le texte de financement de la Sécurité sociale 2 mots suffisent, manque d'ambition et et on ressent un immense ce décalage entre les attentes de notre société pour le grand âge, exprimer de multiples façons et la réalité de ce budget bien sûr quelques dispositions vont néanmoins dans le bon sens, je pense notamment au renforcement du contrôle financier, des Ephad et leur groupe et je salue particulièrement Bernard Bonne, je pense aussi à l'introduction d'un accompagnement au lien social pour les personnes âgées dépendantes jusqu'à deux heures, manière de reconnaître les vertus de l'attention, au-delà du seul soin physiologique, mais ces dispositions avec la poursuite de la refonte tarifaire des soins à domicile ne changeront pas le paysage de la perte d'autonomie, loin de là, le rapporteur Philippe Moulier ne porte pas une analyse différente de la mienne et je sais très attaché, lui aussi, à l'examen d'une vraie grande loi au grand âge et à l'autonomie, le chantier majeur toujours repoussé par le gouvernement reste la convergence des politiques de l'âge et du handicap pour mettre fin aux injustices, face à des incapacités similaire mais survenue à différentes périodes de la vie, les amendements socialistes, par exemple, la levée des seuils d'âge, la prestation universelle de compensation ont été jugées irrecevables dans ce PLFSS et cela rend encore plus nécessaire le besoin d'un texte d'ambition dans ce domaine au delà des missions de cette branche, nous ne pouvons pas passer sous silence la situation alarmante du médico-social, ces métiers peinent à attirer, on y rencontre toujours des personnels exclus du Ségur les aides-soignantes si épuise plus que les travailleurs du BTP, c'est la Cour des comptes, qui souligne qu'il le souligne et qui note qu'une hausse des effectifs serait bénéfique pour le budget de la branche accidents du travail quand même ah cela votre intention d'embaucher 3000 postes cette année, on n'est pas dans une trajectoire de 50000 dans le quinquennat surprend et ne suscite que de la déception, cela représente à peine un demi-poste par iPad à ses besoins criants, s'ajoute désormais la prise en compte de l'inflation, les établissements alerte sur le coup des fluides et votre gouvernement ne pourra pas s'en sortir en proposant de mettre un pull à col roulé à toutes les personnes âgées de nos iPad il y aura pas assez de personnel pour cela les socialistes prennent la mesure de ces enjeux, nous savons qu'il faut augmenter la part des dépenses publiques et nous proposons d'y consacrer des contributions nouvelles comme celle assise sur les dividendes ou sur les bénéfices des Epad privé avec ses moyens nouveaux, nous avons pour objectif de remédier au manque, au manque de place aux délais insupportables, non il n'est pas normal en France d'être sur une liste d'attente pour rentrer en foyer d'accueil médicalisé, ni de devoir patienter 2 ans pour être suivis en centres médico-psychologiques, les soignants s'épuise les aidants désespère les familles attendent agissons. Et chers collègues. La parole est maintenant Madame Jocelyne Guidez pour lui six minutes pour le groupe Union centriste. Monsieur le président, mais mesdames et messieurs les ministres, madame la rapporteure, madame la présidente, mes chers collègues, je souhaiterais d'aborder la 5ème, branche de la Sécurité sociale pour répondre aux besoins croissants de financement, l'objectif de dépense de la branche de l'autonomie, pour 2023 s'élève à 37 virgule 3 milliards d'euros, en augmentation de 5,3 % par rapport à l'année précédente, je tiens à souligner 2 points importants : prévention et vieillir à domicile, d'abord le Plfss pour 2023 accorde une importance particulière à une meilleure prévention avec la mise en place de rendez vous de prévention à certains âges clés de la vie, sans pour autant le rendre obligatoire chez adultes de 60 65 ans, ce rendez-vous permettra de prévenir les malades chroniques, les troupes de vision les fragilités ou la perte d'autonomie, j'ai déposé un amendement visant à repérer les aidants lors de ce rendez-vous et de prévenir les conséquences de la situation des dents sur leur état de santé ensuite le Plfss pour 2023 donne priorité aux vieillir à domicile le plus longtemps possible pour les personnes âgées en perte d'autonomie vivre ces Vié vieillir, rien de plus, écrivez Simone de Beauvoir dans l'inviter, rappelons que 90 % des Français souhaitent vieillir et être accompagnées dans leur vieillissement ou leur handicap à domicile afin de répondre à cette attente de la société civile, quelques mesures phares ont été prises, l'article 33 vise à sécuriser la réforme de la tarification des services de soins infirmiers à domicile, qui devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2023 aussi 4000 places supplémentaires seront créées, l'article 34 permet au département de compléter, voire de dépasser le plafond des plans d'aide personnalisée à l'autonomie par 2 heures d'accompagnement et de temps social lorsque cela est nécessaire, même si cette mesure représente une avancée importante et va dans l'intérêt des professionnels ainsi que des personnes âgées, les sénateur Union centriste regrette profondément son périmètre restreint uniquement aux bénéficiaires de la pas excluant de facto les bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap, par ailleurs, les plans d'aide actuellement des bénéficiaires de la pas ne permettant pas de répondant tout ou partie aux gestes de la vie quotidienne dont ils ont besoin, il est à craindre que ces heures ne se limite qu'à répondre à des besoins vitaux pour les personnes âgées, au détriment des heures de lien social, pourtant nécessaire, par conséquent, nous nous interrogeons sur la soutenabilité de son financement par les départements, malgré les besoins grandissants de la population d'avoir recours aux services à la personne, le secteur à forte intensité de main d'oeuvre est confrontée à de vives tensions en recrutement sur l'ensemble des métiers en ce sens un 1000000 d'emplois sont à pourvoir d'ici à 2030, toutefois, le Plfss pour 2023 ne contient aucune mesure a application immédiate pour ce secteur, le texte présente des éléments positifs comme le bouclier inflation et le bouclier énergie il faudra élargir le bouclier énergie au service à domicile pour lesquels les factures d'essence pèse lourdement, surtout dans les territoires ruraux pour améliorer la prise en charge des personnes âgées dans les EPHAD ce projet de loi prévoit plusieurs mesures revalorisation salariale actualisation des coupes patos déploiement de Centre de ressources territoriaux, la simplification des modalités de financement de l'habitat inclusif, l'aide à la vie partagée est une bonne solution qui retardera les entrées dans les EPHAD par ailleurs les Epad vont bénéficier de 3000 aides-soignants et infirmiers supplémentaires en 2023, même si ces annonces vont dans le bon sens, une réflexion sur les problèmes rencontrés par le secteur s'avère nécessaire attractivité formation VAE postes vacants, comment donner envie à des femmes il et à a des hommes de s'engager dans des services d'aide à domicile, de devenir auxiliaire de vie ou infirmiers en pratique avancée ce spécialisé en gériatrie, nous saluons enfin l'inscription du bien vieillir dans le conseiller national de la refondation adapter la société au vieillissement promouvoir promouvoir la citoyenneté des personnes âgées et le lien social, revaloriser des métiers sont les 3 axes du CNR dédié à la thématique du bien vieillir 10 ateliers de concertation sont prévues dans 10 départements de métropole et d'outre-mer, la feuille de route, issu de la concertation sera présenté en mai 2023, je profite de cette occasion pour mettre l'accent sur la participation des aidants ah ces échanges et la nécessité de l'amélioration des mesures en faveur du répit qui joue un rôle important dans la lutte contre l'isolement social des personnes âgées ou handicapées en ce qui concerne les aidant les articles 34 bis et ter du PLFSS 2023, que le gouvernement a choisi de retenir en faisant usage usage du 49 3, traits de l'élargissement de la durée de l'indemnisation du congé proche aidant ainsi que de l'identification des moyens d'élargir l'allocation journalière du proche aidant aux aidants des personnes malades du cancer, le gouvernement propose de nous remettre des rapports sur ce sujet, je soutiendrai leur maintien dans le texte, sachant que moi-même j'ai demandé depuis plusieurs années, l'article 35 ter, issu d'un amendement ouvre une expérimentation permettant la création d'un véritable parcours d'accompagnement harmoniser des aidants familiaux qui pourrait notamment passer par la prise en charge d'une consultation médicale spécifique rappelons aussi qu'une politique de l'autonomie ne se réduit pas au grand âge au bien vieillir sur le Champ du handicap le PLFSS encourage à transformation des établissements médico-sociaux et promeut les démarche inclusive, nous nous réjouissons de l'augmentation des moyens budgétaires, près de 70 millions d'euros destinés à développer l'offre pour le public, atteint de troubles du spectre de l'autisme, je préférerais parler de trouble du neuro-développement afin de mieux prendre en charge de TDAH et les l'article de 33 terre organise la revalorisation annuelle du tarif plancher qui passera à 23 euros en 2023, l'article 35 bis issu d'un amendement du gouvernement : créer un parcours de rééducation et de réévaluation des enfants en situation de polyhandicap ou de paralysie cérébrale enfin nous regrettons l'absence de présentation par le gouvernement d'une loi grand âge et le manque de projection pluriannuelle indispensable pour relever les défis de cette branche, chers collègues, le secteur médico-social souffrent du contexte de l'inflation et de la crise du recrutement, les oubliées du Ségur de la santé mettent en cause une forte inégalité de traitement, le temps des constats et des propositions est révolu, il est l'heure d'élargir sur le terrain, de mettre en place un plan d'action des dispositifs d'urgence et des modalités concrètes, je vous remercie de votre attention.

Monsieur le président, Mesdames les Ministres Monsieur le Ministre Mesdames les rapporteurs, messieurs les rapporteurs, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, notre système de santé vit depuis quelques années une crise sans précédent alors qu'au 20ème siècle, il faisait figure de référence mondiale, nous devons constater désormais son inadaptation totale face aux défis de la transition écologique de la transition démographique de la transition technologique, les différentes réformes mises en place depuis quelques années, quelques dizaines d'années n'ont pas permis de reconstruire notre système de santé à la hauteur de ces enjeux, malgré la bonne volonté de chacun de leurs auteurs le PLFSS pour l'année 2023 Monsieur le Ministre, est, à l'exemple des précédents, il ne présente aucune réforme majeure, ils modifient à la marge les modalités d'exercice de certains professionnels de santé et continue de mélanger les genres Laurent de financement et loi d'organisation de la santé sur le territoire national, c'est évidemment la meilleure façon d'entretenir la confusion on suce cette fois l'application du 49 3 mettent en doute dans mon esprit, la volonté du gouvernement de respecter la légitimité du Parlement, j'étais naïvement persuadé qu'avec cette nouvelle mandature et avec le constat que nous faisons tous vous alliez présenter un projet qui aurait remis la santé sur les rails, pourquoi ne pas avoir eu la volonté dès ce Plfss de refonder la gouvernance de la santé, en proposant par exemple une loi de programmation sanitaire sur la durée du mandat présidentiel, pourquoi ne pas donner ne serait-ce qu'un signe de votre volonté d'avoir une stratégie de santé fondée sur l'évaluation des besoins de santé et d'objectifs de santé sur 5 ans, pourquoi ne pas développer une vraie politique de gouvernance autonome démocratique de l'hôpital, à la demande du président Larché, fait des propositions au président de la République, propositions qui sont restées lettre morte, pourquoi ne pas marquer votre volonté de mettre en place une vraie démocratie sociale et sanitaire au Centre du fonctionnement de l'hôpital et rééquilibrer le management entre la médecine et l'administration, pourquoi ne pas permettre à la mise en place des patients experts qui apporterait aux soignants, l'expertise des malades, pourquoi ne pas assurer aux professionnels libéraux qui soit garant l'émission territorial de santé, pourquoi ne pas proposer une restructuration de la permanence des soins ambulatoires, afin de garantir la pertinence des urgences hospitalières, pourquoi ne pas réviser les ordonnances Debré pour permettre un meilleur ancrage territorial des hôpitaux je pourrais Monsieur le Ministre, continuer la liste des pourquoi, mais j'entends votre réponse, tout cela sera discuté dans le cadre du Conseil national de la refondation or monsieur le ministre, il y a urgence, et les conclusions de ce conseil n'interviendront que l'an prochain, la mise en place de loi qui Dieu suivront nécessiteront des mois et des mois de mise en forme et nous aurons encore perdu un ou 2 ans, et vous serez contraints, une fois encore de mettre des rustines, c'est le cas actuellement pour la pédiatrie, j'aimerais revenir sur un point plus particulier le financement notre modèle solidaire impose à un financement solidaire, c'est-à-dire dont les ressources et les dispenses respecte le caractère solidaire payer selon ses moyens, recevoir selon ses besoins, cette règle s'applique pour la sécurité sociale mais pas pour les assureurs privés, pratiquement tous les pays développés, qui dispose d'un modèle universel ont un payeur unique de type solidaire, ce système est garant de la liberté des acteurs et de l'indépendance professionnelle des soignants,

pas tous, en particulier les indépendants défavorable pour les inactifs, en particulier les retraités dans les faits, seul le financeur public supporte le vrai risque, seuls 2 financeurs publics garantit le libre choix de son professionnel de santé et l'indépendance professionnelle des soignants, on le voit dans la mise en place des réseaux en matière d'optique ou de certains soins de certains centres de santé dentaire, la liste serait longue, mais nous pouvons constater avec le financement assuranciel privé une diminution de l'équité d'accès aux prestations de santé il serait nécessaire, selon que l'on revoie complètement le système de financement de la santé, à l'instar d'autres pays en Europe, les assurances complémentaires devrait devenir supplémentaires et chacun d'entre nous devrait savoir combien coûte la santé, ce serait d'ailleurs une façon pour le Parlement de fixer chaque année, le tarif de base des organismes complémentaires de santé si j'en reviens au PLFSS telle qui s'impose à nous, celui-ci fait état d'une nette amélioration des comptes avec un déficit à 7 3 milliards d'euros, contre près de 18 milliards en 2022 premières constatations : combien de temps notre système peut-il vivre encore avec de tels déficits 2ème constatation, le Haut Conseil de la santé publique, a émis des doutes sur la sincérité de la de ce Plfss puisque celui-ci s'appuie sur des prévisions macroéconomiques excessivement optimiste avec une surestimation des recettes pour 2023 quant aux dépenses, elles me semblent sous-estimer, surtout au niveau de l'Ondam, ville qui enregistre une augmentation de 0,5 point par rapport à l'Ondam, ville d'avant Covid alors qu'à cette époque il n'y avait pratiquement aucune inflation j'espère aussi que l'estimation des dépenses Covid seront vrai et qu'elles ne seront pas sous-évaluer les on voit bien que d'autres épidémies, arrive l'exemple de la bronchiolite montre à quel point nous avons l'obligation de réussir cette fois les réformes nécessaires, je ne voudrais pas rentrer dans le détail de ce Plfss nous aurons toute cette semaine pour nous exprimer sur les différents articles de ce projet de loi sanctionné par le 49 3 je voudrais simplement revenir c'est la branche famille, si mes souvenirs sont bons, chaque branche a été créé indépendamment des autres branches chaque branche à sa fonction propre et doit occuper intégralement cette fonction depuis des années au nom de je ne sais quel principe des différents gouvernements, quelle que soit leur tendance politique ont ponctionné allègrement la branche excédentaire AT-MP cette fois vous aller plus loin encore en profitant des excédents de la branche famille pour imposer à celle-ci, le remboursement de congé maternité, soit 2 milliards d'euros qui restent évidemment insuffisant pour équilibrer les comptes de la branche maladie, pourquoi monsieur le Ministre, avec ces excédents de ne pas avoir relancé la politique de natalité depuis 2014, les familles ont subi les modulation des allocations familiales dont l'effet cumulé atteint 4 milliards d'euros depuis 2014 la suppression du complément du libre choix d'activité majorer la modulation de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, la fameuse page l'alignement du montant du plafond de l'allocation de base du cours sur le complément familial, il y avait, vous le voyez beaucoup à faire pour améliorer la politique de natalité, je viens de vous exprimer mon désenchantement et mon angoisse de voir notre système devenir obsolète forme faute faute pardon de réforme en profondeur au moment du mouvement des Gilets jaunes, j'avais dit à la ministre, Agnès Buzyn, qu'il fallait éviter le mouvement des Gilets bleu et des blouses blanches. La crise Covid est passé par là, mais la réalité nous rejoint à nouveau, il est grand temps de réagir car comme chanter, comme le chantait pardon Barbara le temps qui passe ne se rattrape pas le temps perdu ne se rattrape plus. La parole est maintenant à madame la présidente, Laurence Rossignol pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour 3 minutes. Monsieur le président, Mesdames et messieurs, et monsieur le Ministre, chers collègues, je regrette que le ministre chargé des solidarités ne soit. Tu dans l'hémicycle pour le moment où on parle aussi de la solidarité, le PLFSS ce n'est pas que que l'assurance maladie et en particulier je vais poursuivent ce que a dit mon collègue un instant sur la ponction effectuée sur la branche famille qui est désormais non seulement à l'équilibre, mais excédentaire, ce qui donne des marges considérables au gouvernement pour ré-initier une politique familiale adaptée moderne qu'on compatibles et conciliant la volonté des familles et en fait avec cet excédent de la branche famille, vous faites un petit jeu comptable dont j'imagine bien qu'il a été, dans les cerveaux de Bercy puisque Bercy a la tutelle aussi sur le PLFSS et le jour où nous avons accepté ça, nous avons fait une énorme faute Bercy ce PLFSS ben où prendre l'argent pour le PLFSS et qu'elle prendra la famille ceci dit c'est pas tout à fait neutre parce que, comme Bercy réfléchissent pas comme les ministres de la solidarité, solidarité ou de la santé, c'est pas tout à fait neutre parce que ça a du sens que de ne plus prendre en charge au titre de l'assurance maladie des années petit journalière et de les transférer sur la branche famille, la famille, la politique familiale est une politique qui est fondé sur le choix les familles ont le choix : le choix du mode de garde, le choix de prendre des congés familiaux la préparer le c'est le choix

mais plutôt au-delà de l'hémicycle, les associations familiales, c'est que le congé les Ziggy post-accouchement, ce n'est pas un congé pour s'occuper de l'enfant, c'est un congé qui a rendu nécessaire par la santé de la mère et la protection maternelle et l'aligné sur le congé de paternité en terme de financement c'est le faire rentrer dans ses congés à option parce que l'étape suivante, je l'imagine bien on demandera au papa et à la maman de choisir lequel des deux prend le congé post-accouchement je voulais attirer votre attention là-dessus 2ème sujet dont je veux paraît en très peu de temps, c'est la déconjugalisation de l'allocation de soutien familial, je vais faire court, j'ai aujourd'hui une mère de famille veufs 2 enfants mille euros par mois, hein, pas son invalidité plus 300 euros de revenus qui se fait, qui se voit demander par la CAF 5 euros de trop perçu de son allocation de soutien familial parce que elle a un homme dans sa vie qui lui-même gagne le SMIC et lui-même à un enfant à charge et la caisse de location familial considère que cet homme est supposée prendre en charge les enfants de cette femme seule déconjugaliser l'allocation de soutien familial, c'est une exigence pour les familles monoparentales, pour les mères pour la lutte contre leur solitude et tout simplement pour qu'elles aient un niveau de vie correcte, oui, oui, Monsieur le Ministre, je vois que vous que vous c'est normal vous croyez n'était pas le dossier, mais c'est comme ça, quand une mère de famille monoparentale, à une nouvelle relation amoureuse, on lui supprime son allocation de soutien familial, au motif qu'elle n'est plus seul et que le nouvel homme de sa vie supposée de financer l'entretien de ses enfants, mais ce n'est pas normal comme la présidente. Bien. Je sais pas qui commence, c'est vous, Monsieur le Ministre, allez-y. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs Madame la rapporteure générale, madame la présidente, je ne reviendrai pas sur l'ensemble des remarques qui ont été faites, j'aurai l'occasion pendant les débats de revenir si vous le souhaitez, point par point. Pour compléter des informations je tenais toutefois à dire que je suis sensible à ce que la rapporteur général a exposé concernant la nécessaire rectifications de le dames 2022 cette rectification avait été proposé dans le texte initial qui n'avait pas été retenue par l'Assemblée nationale, je suis de de toute évidence, favorables à ce rétablissement, élément essentiel pour la crédibilité de ce Plfss et qui garantira un financement nécessaires pour le système de santé en 2022 toutefois, pour aller plus loin, le gouvernement propose un sous-amendement pour aller au-delà de ce temple rétablissement proposée par la rapporteuse générale et ajouté encore 600 millions d'euros sous objectifs d'établissements de santé et donc à l'Ondam 2022 dans son ensemble, il s'agit de financer les engagements pris pour assurer le bon fonctionnement des établissements de santé, dans cette période actuelle de crise d'épidémies hivernales de financer une partie des engagements des dernières annonces que j'ai pu faire concernant les établissements en tension et particulièrement les services de pédiatrie. Que j'assure là encore comme je les vois régulièrement de mon soutien le plus entier face à cette crise difficile il faut certes faire un traitement symptomatique immédiat mais nous démarrons également avec eux les travaux sur le traitement de fond qui aboutira, comme je l'avais annoncé aux assises de la santé de l'enfant au printemps et qui proposera une feuille de route pour les années à venir autour de la santé de l'enfant ces crédits supplémentaires permettront notamment de soutenir financièrement les agents qui travaillent la nuit et en soins critiques, en particulier pour les pierres et les aides Pierre. Cette rectification de l'Ondam établissements permettra aussi de solvabiliser les établissements de santé qui ont déployé les mesures de cet été de la mission flash, en particulier les heures supplémentaires et le temps additionnel la rectification de l'Ondam 2022 est ainsi porté à 9,7 milliards par rapport au montant voté dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 par cette décision, le gouvernement matérialise à nouveau sa détermination à consacrer tous les moyens nécessaires au bon fonctionnement des établissements de santé. Merci, monsieur le Ministre, Madame la Ministre. Merci monsieur le président, je serai pas très long, mais vous avez été nombreux et notamment Madame la rapporteure à questionner la stratégie économique, macro-économique qui sous-tend ce PLFSS et qui a fait l'objet de plusieurs remarques, je souhaite préciser premièrement que le Haut conseil aux finances publiques a effectivement rendu un avis positif sur le scénario macroéconomique des textes financiers cet Automne, les prévisions de croissance et d'inflation ont été jugés et j'emploie leur mot crédible tout comme la prévision d'inflation en 2023 la prévision de croissance pour 23 a été jugée un peu élevée mais le Haut Conseil relève bien lui aussi la forte incertitude qui cours cette prévision et qui concerne tous les pays développés, la prévision de masse salariale pour 2023, en hausse de 5 % % a également été jugé plausible, c'est donc un tableau plutôt nuancé et cet été déjà, on avait eu ce débat qui me semble important, et le Haut Conseil jugeait un peu élevé pour le coup, la prévision de croissance à 2,5 % pour 2022 aujourd'hui l'Insee nous dit qu'avant même de comptabiliser le quatrième trimestre, l'acquis de croissance pour 2022 s'élève déjà à 2,5 je rappelle aussi que la France est sortie un peu plus rapidement de la crise que ses voisins, retrouvons défunt 21, un niveau de production d'avant crise. Tout ça, et notamment le quoi qu'il en coûte, a directement contribué à maintenir l'investissement à un niveau toujours dynamique, je veux partager avec vous que l'investissement des entreprises, selon la dernière note de conjoncture, qui vient de sortir de l'Insee, en date du 28 octobre dernier l'investissement des entreprises devrait croître d'au moins de en 2022, le climat des affaires, quant à lui, mesuré également par l'Insee, comme vous le savez, reste un peu supérieur à la norme avec un niveau de 100 de contre 100 en moyenne, les créations d'emplois s'élève à 220000 au 1er semestre comme je l'ai rappelé vous dire que les textes financiers qui vous sont soumis cet Automne que soit le PLF le PLFR ou encore le PLFSS comporte des mesures justement pour atteindre le 1 % de croissance en 2023, avec notamment la poursuite d'un soutien vigoureux aux entreprises, mais aussi aux collectivités territoriales face aux effets de l'inflation, ce soutien s'est illustré, vous le savez, d'abord par l'adoption d'un filet de sécurité de 430 millions d'euros en 22 de un virgule d'euros en 23 pour les collectivités, mais aussi, et vous le savez, par la poursuite du bouclier tarifaire pour les ménages qui représentent une masse financière de 100 milliards d'euros et qui permettra d'éviter une dépense allant de 160 à 175 euros par mois et par foyer français au total, mesdames, messieurs les sénateurs, sans être trop longue, je voudrais juste rappeler que l'économie française, malgré les difficultés continuent au moment où on se parle, a résisté, que c'est à l'aune de ces hypothèses et de cette réalité que nous avons fondé les éléments du PLFSS ça n'est ni une vision optimiste, encore moins une vision démesurément optimistes ni une vision d'ailleurs pessimiste de la conjoncture s'est semble-t-il bien l'état de notre pays et c'est donc à l'aune de ce tableau macroéconomique que les grands arbitrages et les grands équilibres du PLFSS qui vous ont été présentés, je vous remercie. Merci madame la ministre, madame la présidente. à peine à la moitié des amendements déposés en examen c'est pas sympa mais ce sera une heure et après on laissera un petit peu de temps pour aller dîner et on continuera demain bien aimable, madame la présidente. Bien, je vais suspendre la séance, elle sera reprise à 21 heures 30 pour la suite de l'examen de ce texte, la séance est suspendue.